Il y a un an, presque jour pour jour, ce mot terrible, que l'on croyait banni du continent européen, a résonné de nouveau en Europe. Il ne s'agit pas d'une guerre allégorique, de celles que l'on déclare de façon galvaudée dans une situation d'adversité. Il s'agit bien d'une guerre réelle, d'une guerre d'agression, dans toute sa brutalité. À vrai dire, la guerre n'était pas chose nouvelle en ce 24 février 2022. Votre peuple, monsieur le président de la Rada, connaît la guerre depuis 2014, depuis l'agression de la Russie et l'occupation d'une partie de l'Ukraine, neuf années déjà, même si ces derniers mois furent d'une intensité rarement égalée. Ce qui a changé, à partir du 24 février 2022, ce fut la mobilisation, inédite, des soutiens de l'Ukraine dans le monde, au sein de l'Union européenne et en France, depuis le sommet de l'État jusqu'aux simples citoyens, sans sans oublier nos collectivités territoriales. En effet, il faut le reconnaître avec lucidité : en 2014 et dans les années qui suivirent, à l'exception des Ukrainiens, agressés, et de quelques pays européens, nous n'avions pas pris, collectivement, la véritable mesure de ce qui se produisait sur le sol de l'Ukraine et du danger représenté par l'impérialisme russe. Ce passé, fait d'irrésolutions, est désormais derrière nous. Votre cause est devenue la nôtre, parce que nous savons que l'Union européenne ne sera pas en paix si la Russie est victorieuse en Ukraine. Nous n'avons qu'un objectif, et un seul : que demain l'Ukraine soit libérée

ont constitué un tournant supplémentaire dans la détermination collective à vous soutenir. Cet engagement est appelé à perdurer et à ne pas faiblir. Nous formons le voeu que la France, dans le cadre d'une aide militaire cohérente et concertée avec ses partenaires, continue d'apporter une contribution substantielle à votre système de défense, pour mieux protéger les populations civiles et vos installations stratégiques, et pour vous aider à résister et à reconquérir le territoire de l'Ukraine internationalement reconnu. « Risque d'escalade », entend-on ? Cette interrogation est légitime. Mais quelle est l'autre solution laissée par la Russie ? Ce n'est pas l'Ukraine qui nous contraint à livrer toujours plus de matériel, c'est la poursuite de l'agression et des exactions russes qui nous l'imposent ! La France et l'Union européenne, à la différence de l'Ukraine, ne sont pas en guerre

l'avantage stratégique. Nous devons l'y aider. Monsieur le président, il y a six mois, en juillet 2022, vous m'aviez accueilli, ainsi qu'une délégation de sénateurs, dans l'enceinte de la Rada et vous m'aviez donné l'occasion de prononcer un discours en séance plénière, devant tous les parlementaires. Mes chers collègues, peut-on se figurer un parlement réuni régulièrement sous la menace permanente des alertes à l'approche de missiles destructeurs ? Tel est le quotidien de nos collègues parlementaires de la Rada. En résistant, les Ukrainiens démontrent que l'héroïsme n'est pas la vertu des causes désespérées. Je souhaite, mes chers collègues, que nous nous levions pour rendre hommage au courage de nos collègues parlementaires de la Rada, ainsi qu'à celui de tous les Ukrainiens, et que nous les applaudissions.

Le 7 février prochain, le Sénat débattra d'un projet de résolution en soutien à votre pays qui dépasse les clivages politiques et qui, je l'espère, recueillera les plus larges suffrages. Le projet de résolution ne se contente pas de répéter les résolutions précédentes : il fait sien le plan de paix présenté par le président Zelensky lors du sommet du G20, le 15 novembre 2022 : la souveraineté de l'Ukraine sur l'ensemble de son territoire n'est pas négociable. La Crimée ou le Donbass n'ont qu'une vocation : être ukrainiens. Surtout, le projet de résolution du Sénat insiste sur l'impératif de justice, afin que les criminels qui, au nom de la Russie, commettent des exactions et des crimes de guerre, persécutent et exécutent des civils sachent qu'ils ne bénéficieront d'aucune impunité, parce que l'impunité ouvre la voie aux plus grands crimes et à la manipulation de l'histoire. En témoigne la négation persistante par les autorités russes de ce qu'il conviendrait de reconnaître comme le génocide de l'Holodomor, en 1932 et 1933. Monsieur le président de la Rada de l'Ukraine, mes chers collègues, le moment que nous partageons aujourd'hui est exceptionnel, sinon inédit. Si le président Zelensky s'est exprimé le 23 mars 2022 en visioconférence devant le parlement français, jamais l'hémicycle du Sénat n'a accueilli le président du parlement d'un pays en guerre.

Seuls le président du Bundesrat allemand et la présidente du Parlement européen ont eu, par le passé, cette occasion. C'est dire la dimension européenne qui est conférée à cette tribune. C'est dire le degré d'amitié et de confiance que le Sénat témoigne à la Rada et à son président. Oui, vraiment, vive l'Ukraine, vive la République et vive la France ! La parole est

les paroles de l'Ukraine en proie aux flammes. Depuis cette haute tribune du Sénat parleront aujourd'hui des millions d'Ukrainiens qui vivent

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes-vous demandé pourquoi on nous tue ? On nous tue uniquement parce que, tout comme vous, nous aimons notre terre ; parce que, tout comme vous,

toutes les armes disponibles : les missiles balistiques, les drones kamikazes ; on nous tue par le froid et l'obscurité, en détruisant les infrastructures énergétiques critiques. Vous êtes-vous Vous êtes-vous demandé qui nous tue ? Celui qui, sous couvert d'une « opération militaire spéciale », a lancé cette invasion à grande échelle, celui qui rêve de restaurer l'empire russe ou l'Union soviétique, celui qui fait fi du droit international international et des normes de coexistence pacifique. C'est sur son ordre que nous sommes tués par ceux qui, hier encore, nous juraient être nos frères. « L'opération militaire spéciale » en Ukraine,

La bête se présente aujourd'hui comme un agneau, mais elle aspire toujours à tuer et à s'emparer de nouveaux territoires. Chers amis, un grand penseur français, René Descartes, a dit en son temps

d'obtenir des avions, des blindés lourds et des moyens de défense anti-aérienne et anti-missiles, pour avoir la supériorité au sol et fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine.

il n'y a pas de mots assez forts pour vous exprimer notre reconnaissance d'avoir accueilli en France plus de 100 000 de nos concitoyens, qui sont aussi de futurs citoyens de l'Union européenne. Je vous remercie

j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles de notre assemblée : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe Les Républicains. Ma question à Mme la Première ministre. Madame la Première ministre, depuis une semaine, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites paralyse notre pays, ce qui provoque une nouvelle fois l'exaspération de nos compatriotes dépendant des transports publics. Comme d'habitude, ce sont les Français les plus fragiles qui sont pénalisés, ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre des jours de congé ou de télétravailler et qui n'ont d'autre solution de transport que le train, le bus ou le métro. Il n'est pas acceptable qu'une minorité de Français prenne ainsi en otage les salariés qui veulent travailler, mais aussi nos artisans et commerçants déjà lourdement affectés par les crises sanitaire et énergétique. Si le droit de grève est garanti par la Constitution, il n'est pas pour autant un droit de blocage de tout un pays. Bien que la loi de 2007 ait organisé l'information des usagers en cas de grève, elle n'a pas permis d'aboutir à un service minimum garanti. C'est ce qui a conduit le Sénat à adopter, le 4 février 2020, une proposition de loi de notre collègue Bruno Retailleau, qui permet enfin de limiter le droit de grève si cela se révèle nécessaire pour garantir un service minimal. Madame la Première ministre, ne croyez-vous pas qu'il est grand temps de reprendre ce texte à votre compte et de le faire adopter dans les meilleurs délais ?

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes nombreux sur toutes les travées à avoir soutenu la révolution en Iran, notamment en parrainant des prisonniers

Les musulmans se vengeront. Vous arrêterez les assaillants, mais les morts, eux, ne reviendront pas. » Quant au ministre des affaires étrangères iranien, il a déclaré : « Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les limites. » Il ne se demande pas en revanche si l'Iran a dépassé les siennes ! J'ajoute que les gardiens de la révolution ont leur milice à l'étranger et une branche armée capable d'agir partout dans le monde.

la situation risque de dégénérer. Notre sécurité est clairement menacée. Dans ces conditions, madame la secrétaire d'État, ma question est simple : quelles mesures entendez-vous prendre ou avez-vous déjà prises pour protéger les Français ?

Nous répondons en Européens, en prévoyant des sanctions pour accompagner les revendications légitimes des Iraniennes et des Iraniens et garantir qu'il n'y aura aucune impunité pour les auteurs de la répression et de ces menaces. Comme vous le savez, quatre trains de sanctions

Les sanctions prises à l'encontre de personnalités européennes participent du même aveuglement que celui dont fait preuve le régime iranien lorsqu'il s'enferme dans le déni ou la rhétorique complotiste et mène une politique scandaleuse d'otages d'État.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Il y vantait les bienfaits de la réforme des retraites de ce gouvernement, qui, pourtant, ne cesse de perdre en popularité, même en son sein. De très nombreux fonctionnaires ont été choqués de recevoir sur leur adresse mail personnelle, la direction générale des finances publiques, une telle vidéo de propagande. Monsieur le ministre, estimez-vous qu'il est démocratiquement légitime et

les spécificités du régime de retraite de la fonction publique, c'est-à-dire un mode de calcul des pensions sur les six derniers mois d'activité, en précisant d'emblée que le taux de remplacement n'est pas plus élevé dans le système public que dans le système privé, ainsi que le bénéfice de la catégorie active.

cela se voit dans la vidéo, tout comme dans les déclarations d'Élisabeth Borne, qui nous explique que les 64 ans ne sont pas négociables. Mais écoutez l'opinion publique ! La rue vous a parlé encore hier. Des millions de personnes sont sorties manifester contre votre réforme injuste. Le message est clair,

La parole est à M. Michel Dagbert, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Au-delà, c'est l'ensemble des métiers du social et du médico-social, qu'il s'agisse de la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des adultes qui connaissent des difficultés sociales ou de la protection de l'enfance qui

prennent parfois la forme d'injonctions émanant de leurs employeurs privés ou semi-publics. Cette double exigence explique en grande partie la perte d'attractivité de ces emplois et les difficultés de recrutement qu'ils rencontrent actuellement. À titre d'exemple, les instituts de formation nous indiquent que 30 % des étudiants arrêtent avant la fin de leur cursus. Je vous sais, monsieur le ministre, très attentif aux travaux et préconisations émises par le Haut Conseil du travail social dans ses différents rapports. Je ne doute pas de l'intérêt que vous portez à la fois aux professionnels concernés et aux personnes dont ils ont la charge. Pourriez-vous dès lors nous indiquer les dispositions que vous comptez prendre

et Républicain. Madame la Première ministre, pour la quatrième semaine consécutive, nous vous interrogeons sur la réforme des retraites. Et je crains que, pour la quatrième fois consécutive, vous ne persistiez

défendez cette réforme en l'inscrivant dans une démarche de défense du modèle social français. Mme Brigitte Macron, pour sa part, a affirmé qu'elle était nécessaire pour assurer une retraite aux jeunes. Pendant ce temps, le Président de la République la juge « indispensable quand on se compare à l'Europe ». Bref, mes chers collègues : une réforme idéale, la mère de toutes les réformes ! Alors, que demande le peuple ? Eh bien, le peuple vous a donné hier dans la rue, toutes générations et tous territoires confondus, une éclatante réponse. Il ne veut pas de votre réforme, de ce nouvel impôt sur la vie que vous défendez avec obstination, quoi qu'il en coûte. Ce que nous savons, c'est que le « rendement financier »- pour reprendre votre expression, madame la Première ministre -de votre réforme sert à faire des économies sur le dos des ouvriers et des employés, qu'ils soient issus des classes populaires ou des classes moyennes. faire ces économies ailleurs et éviter de prendre aux Français les plus modestes ? Ce que nous savons, c'est que vous voulez offrir au Président de la République « sa » grande réforme. J'en suis désolé, mais nous n'avons cure de l'ambition personnelle d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres priorités quand la fracture sociale s'aggrave, quand l'inflation rogne le pouvoir d'achat des petits salaires, quand des étudiants, des salariés pauvres et des personnes âgées font la queue devant les soupes populaires. Écoutez les Français et répondez à ma question : quand retirerez-vous votre réforme des retraites ?

il y a selon moi des principes essentiels en politique : dire la réalité aux Français sans tordre les chiffres, sans vendre d'illusions et sans relayer des contrevérités. Très bien ! Aussi, parlons de faits. Franck Riester ? Aujourd'hui, le nombre d'actifs qui cotisent diminue par rapport au nombre de retraités : c'est un fait. Dans les années 1950, il y avait quatre actifs pour un retraité.

C'est une réalité démographique, qui menace notre système de retraite par répartition. De ce fait, notre système de retraite sera en déficit dans les prochaines années, et ce déficit va s'aggraver. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis ou mon gouvernement qui le décrète : c'est un fait partagé par le Conseil d'orientation des retraites ! Je vous le rappelle : aucun scénario du COR ne prévoit l'équilibre de notre système en 2030. D'ici à dix ans, ce sont près de 150 milliards d'euros de déficit que nous cumulerons et que nous laisserons à notre jeunesse si nous ne faisons rien. raison pour laquelle le Premier président de la Cour des comptes a déclaré la semaine dernière que notre système de retraite n'était pas soutenable en l'état et qu'une réforme était indispensable. Voilà pour les faits, monsieur le président Kanner. maintenant aux conséquences. Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, les organisations syndicales et les différents groupes parlementaires, c'est de l'avenir de notre système de retraite par répartition, en travaillant progressivement plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens. Pas tous ! C'est aussi le choix que des majorités de droite et de gauche ont fait avant nous. Je vous rappelle, monsieur le président Kanner, que vous avez vous-même, avec le parti socialiste, soutenu la réforme de Mme Touraine, qui allait exactement dans le même

... Vous avez changé d'avis, disais-je, et c'est votre droit. Mais que proposez-vous ? Pour financer notre modèle social et pour combler ce déficit, il n'y a que deux autres options. Soit vous voulez baisser les pensions et vous pénaliserez ainsi les petites retraites et les classes moyennes, en les privant du fruit du travail d'une vie, ... Mensonge ! ... soit vous voulez augmenter drastiquement les cotisations et les impôts pesant sur les salaires ou pénalisant les artisans, les TPE, les PME et tous ceux qui font notre vie économique, brisant ainsi la dynamique de l'emploi. Monsieur le président Kanner, puisque nous partageons une volonté commune de vérité, exposez-nous de rechange que vous proposez aux Français : la baisse du pouvoir d'achat ou la hausse du chômage ? Démagogie ! Mesdames, messieurs les sénateurs, notre projet est animé par une seule volonté : assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. Nous portons un projet qui permet le retour à l'équilibre en 2030, en travaillant progressivement plus longtemps. Je mesure ce que cela représente pour de nombreux Français, et je sais que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. C'est pourquoi nous avons veillé à répartir l'effort le plus équitablement possible, notamment en tenant compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui ont un métier difficile.

les plus petites pensions des futurs retraités comme des retraités actuels. Nous pourrions peut-être au moins nous retrouver sur ce point, puisqu'il était défendu par votre candidate à l'élection présidentielle

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

cela ne s'arrêtera pas, non plus, de sitôt. Bien sûr, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires interviennent avec le courage et le dévouement qui les caractérisent. Mais jusqu'à quand et dans quelles conditions ? En effet, l'inflation et la crise énergétique sont passées par là, gelant la capacité d'action de notre sécurité civile.

Au-delà de ces difficultés conjoncturelles majeures, pour lesquelles nous demandons à l'État d'intervenir, nombre d'élus membres des Sdis dressent le constat d'un modèle de financement qui n'est plus adapté aux charges croissantes de nos sapeurs-pompiers. Or, en matière de sécurité civile, tout défaut d'investissement ne pardonne pas. Monsieur le ministre de l'intérieur, « Sauver ou périr », telle est la devise de nos sapeurs-pompiers. Pour aider les Sdis fortement fragilisés, réformer les modes de financement et promouvoir plus de péréquation entre les Sdis au nom de la solidarité nationale,

L'intelligence artificielle peut être un formidable outil si elle est correctement utilisée. Et quoi de mieux que des cours de technologie dès la classe de sixième pour former nos enfants à ces nouvelles technologies Pourtant, vous ne semblez pas être du même avis, monsieur le ministre, puisque, le 12 janvier dernier, vous avez annoncé, par voie de presse, la suppression de la technologie en sixième, au collège. Cette annonce brutale a été un coup de tonnerre pour la communauté enseignante. Cette décision verticale n'a été ni présentée, ni discutée, ni concertée. Elle traduit une méconnaissance totale des enjeux du XXI siècle. En effet, pour réussir la transition écologique qui s'impose à nous, la France a de plus en plus besoin d'une jeunesse ouverte aux sciences et aux technologies. Les méthodes d'apprentissage, propres aux disciplines expérimentales, développent l'esprit critique, stimulent la créativité et contribuent à la lutte contre le décrochage scolaire. Cette suppression serait guidée par des choix budgétaires, sans aucune considération pédagogique. Vous souhaitez renforcer l'accompagnement des élèves en mathématiques et en français, mais sans investir dans l'école de la République. Puisque vous n'avez pas fait de concertation, et afin de susciter votre intérêt pour cette matière, j'ai donc choisi d'interroger ChatGPT pour formuler ma question. Voici sa réponse : « Le Gouvernement peut-il détailler les motivations et les conséquences prévues de la suppression de la technologie en sixième ?

jeunesse. Madame la sénatrice de Marco, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour vous répondre. L'école de la République ne peut laisser de côté un quart et un tiers des élèves de sixième qui ont des difficultés, possiblement insurmontables, en français et en mathématiques. Comme je l'ai annoncé, lors de la rentrée 2023, des sessions de soutien ou d'approfondissement auront lieu dans ces deux disciplines fondamentales

ni suppression de la technologie au collège ni relégation de cette discipline. Au contraire, nous devons faire en sorte que cette discipline soit revalorisée, afin qu'elle suscite des vocations pour le numérique, le numérique, pour les sciences de l'ingénieur et pour la voie professionnelle et qu'elle participe à l'équilibre entre filles et garçons. Concernant les professeurs de technologie, leurs situations personnelles seront préservées et ils bénéficieront, en vue

L'écologie de proximité, l'écologie de l'action, est déterminante pour la réussite de nos objectifs. Nos forces et notre dynamisme pour la transformation se trouvent dans nos territoires. Nos élus locaux sont les acteurs majeurs et les pivots du dispositif. Ils connaissent parfaitement les attentes, les projets et les évolutions de leurs territoires. Pour transformer l'essai, ils doivent être accompagnés d'une offre d'ingénierie solide. C'est décisif pour être en capacité de « délivrer », monsieur le ministre.

flexibilité et stockage, pour créer un circuit court de consommation d'électricité et réduire les coûts de l'énergie. Ce projet d'autoconsommation collective a vocation à hybrider différents types de bâti ; il concerne le privé et le public et, pour ce dernier, à la fois l'État et les collectivités. n'entre dans aucune case. Il a pourtant le mérite de soulever l'enthousiasme de nos concitoyens en zone rurale et, monsieur le ministre, de redonner de l'espérance. Outre qu'elle répond concrètement, selon un mode collaboratif, à des questions très prégnantes, cette initiative auboise n'est qu'un exemple parmi d'autres.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer. En 2022, le nombre de titres de séjour, autorisant à résider et à travailler en France, a augmenté de plus de 17 % par rapport à son Ainsi, plus de 320 000 titres ont été délivrés, contre un peu plus de 277 000 en 2019, qui est la dernière référence significative avant la pandémie. Jamais la France n'a attribué autant de titres de séjour et accueilli autant de demandeurs d'asile, alors qu'elle peine toujours à expulser les illégaux qui vivent sur son territoire. Cette situation, difficilement tenable, témoigne de l'incroyable pression migratoire qui s'exerce sur notre pays. En effet, comme vous le savez, on dénombre près de 700 000 clandestins sur le sol national. Ces chiffres sont en total décalage avec le discours offensif de votre gouvernement sur la question des expulsions de clandestins. Si vous privilégiez la qualité sur la quantité en reconduisant prioritairement les délinquants et les terroristes étrangers sortant de prison, il n'en reste pas moins que les procédures d'éloignement, recensées par vos services, sont au nombre de 19 425 pour l'année 2022. Et ce chiffre reste en deçà de celui d'avant la crise sanitaire sanitaire : M. Castaner avait ordonné presque 24 000 reconductions à la frontière en 2019 ! Résultat, il y a un quart d'expulsions en moins par rapport à 2019, et cela correspond à moins de 3 % du nombre des personnes qui se trouvent en situation irrégulière sur le sol français. La maîtrise des flux migratoires doit imposer de reconduire effectivement les immigrés illégaux, pour accueillir les ayants droit dans les meilleures conditions. Cela suppose des intentions fermes et des actes clairs. Aussi, monsieur le ministre, ma question est simple : qu'attendez-vous pour mettre fin à cette situation insoutenable pour notre pays ?

Vous avez déclaré, monsieur le ministre : « Nous pouvons être fiers d'être le pays au monde le plus ambitieux en matière de lutte contre ces granulés. » Je vous remercie, monsieur le ministre, de reconnaître notre travail parlementaire, puisque c'est grâce à un amendement que j'ai défendu, lors de l'examen de la loi que les entreprises doivent adopter des procédures prévenant la dispersion des granulés. Cependant, monsieur le ministre, l'amendement voté au Sénat était bien plus contraignant, puisqu'il visait

suite, la situation que vous décrivez s'est étendue aux côtes de la Manche et à une partie des côtes flamandes, à l'occasion du week-end, puisque cette fameuse marée blanche a commencé au niveau de la Vendée et de la Loire-Atlantique.

coups et blessures, + 14 % ; cambriolages + 11 % ; vols de véhicules, + 9 %. Avec 879 victimes de crimes en 2022, nous sommes désormais face au niveau le plus élevé depuis trente Ces chiffres ne proviennent ni de ni de. Ce sont les chiffres officiels de votre ministère, et nul ne pourra donc les contester. Cependant, derrière ces chiffres, il y a des réalités. Des Françaises et des Français vivent dans la peur. L'insécurité est devenue une triste réalité, qui n'a cessé de croître pendant les quinquennats d'Emmanuel Macron. Mon département de Lot-et-Garonne, à l'image des autres, souffre cruellement de cette politique. Le quotidien de nos forces de l'ordre est extrêmement difficile manque de moyens humains et de matériel, découragement- le mot est faible -, absence de réponse pénale, voyous qui font la loi partout et qui n'ont peur de rien ni de personne. Oui, les policiers et les gendarmes font ce qu'ils peuvent, mais encore faudrait-il des condamnations fortes. Ah ... Vous ne pouvez pas sans cesse renvoyer la faute sur vos prédécesseurs. L'insécurité, monsieur le ministre, n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un manque de courage et d'une absence de volonté politique. Monsieur le ministre, face à cette délinquance explosive, le Gouvernement est-il vraiment en capacité de protéger les Français ?

choses, monsieur le garde des sceaux, mais ce n'est pas celle des Français. Pierre Dac disait : « Certaines personnes jouent aux échecs, d'autres les collectionnent. » Il est navrant de reconnaître que le Président de la République est davantage collectionneur que joueur.

Cette manoeuvre scelle la volonté de la puissance publique de sauver un groupe privé à la dérive. Une telle opération intervient en réaction à l'un des plus grands scandales sanitaires, déclenché par la parution du livre de Victor Castanet.

quelle est la vision du Gouvernement s'agissant de la dépendance de nos aînés ? Plus précisément, au vu du vieillissement de la population et de l'accroissement des besoins en matière de dépendance, que comptez-vous faire afin d'empêcher que les logiques de marchés et la pression d'actionnaires avides ne l'emportent sur la satisfaction de l'intérêt général ? La parole

la semaine dernière, je répondais à une question de votre collègue, Mme la sénatrice Michelle Meunier, en détaillant ce qui avait été réalisé par l'État depuis

en direction des personnes âgées et d'élaborer une loi sur la dépendance digne de ce nom, d'autre part, d'accélérer et d'amplifier le contrôle sur les établissements à but lucratif. L'argent ne doit pas être l'élément moteur de l'accompagnement de nos aînés. est inacceptable, et je crois nécessaire qu'il y ait une réaction forte de l'État pour protéger nos plus vulnérables. La parole

à la fois pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Permettez-moi aujourd'hui de revenir plus particulièrement sur ses conséquences pour les communes. Celles-ci ont bien entendu engagé, pour la plupart d'entre elles au moins, différents plans de sobriété énergétique dès l'année dernière. Mais, si les effets commencent tout doucement à se faire sentir, ils restent naturellement minimes par rapport à l'impact exorbitant des charges d'énergie sur les budgets Par ailleurs, alors que les communes supportent entièrement les nouveaux prix du gaz, le bouclier tarifaire- pour certaines -, l'amortisseur électricité et le filet de sécurité ne suffisent pas au maintien des équilibres financiers précédents.

Ainsi, il n'est pas rare que, de ce seul fait, l'augmentation des dépenses de fonctionnement d'une année sur l'autre dans la préparation du budget pour 2023 soit de l'ordre de 20 et rende impossible le vote d'un budget à l'équilibre. Monsieur le ministre, il convient de tout faire pour accompagner mieux encore ces collectivités locales en 2023. J'ai, à cet égard, deux propositions à vous Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de prononcer une suspension temporaire, pour 2023, du prélèvement annuel que subissent un grand nombre de communes de notre pays pour insuffisance de logements sociaux, tel que le prévoit l'article 55 de la loi du

alors que les collectivités locales ne peuvent pas récupérer cette taxe. Comment leur éviter cette double peine ? Allez-vous leur faire profiter en retour des sommes ainsi perçues ? La parole est à M. La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Les femmes en sont les premières victimes. Les mères célibataires, dont un tiers sont pauvres, vivent souvent dans des logements précaires et sous-dimensionnés. Pour les Français modestes, et même pour les Français de condition moyenne, le parc locatif privé est totalement inaccessible.

conséquence en est une production HLM au plus bas, avec moins de 85 000 logements construits en 2022, soit une diminution de 30 % par rapport à 2017. Désormais, 2,3 millions de ménages sont en attente d'un logement social.

face au constat de la Fondation Abbé Pierre, toujours plus douloureux chaque année, comptez-vous changer le cap de la politique du logement du Gouvernement ?

pour la réplique. Monsieur le ministre, j'entends vos réponses et je sais l'effort que vous faites. Mais il y a un manque cruel de logement social dans ce pays

En effet, dans une tribune publiée dans le journal, une cinquantaine d'élus animalistes ou écologistes, dont 11 sont membres du conseil municipal de Montpellier, ont mis le feu à la Camargue et à la Petite Camargue. Ils militent pour l'abolition des lâchers de taureaux dans nos rues, la suppression de l'utilisation d'un crochet lors des courses camarguaises, mais aussi l'interdiction des ferrades et de l'escoussure. Nos festivités camarguaises représentent, au-delà d'un enjeu économique certain, une question culturelle importante pour de nombreuses communes dans les départements du Gard, mais aussi de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Avant le grand rassemblement en faveur de nos traditions camarguaises prévu le 11 février prochain à Montpellier, ma question est double.

en 2021, par les sénatrices Catherine Dumas et Marie-Pierre Monier sur le patrimoine culturel immatériel. Tout cela est bien lié à votre intervention, puisque ce patrimoine culturel immatériel comprend les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire, mais aussi tous les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui leur sont associés. Récemment, nous avons obtenu l'inscription des savoir-faire de la baguette de pain. Pour ou contre

Celle-ci évoque nos gardians et nos pêcheurs. Elle incarne trois vertus : la foi, la charité et l'espérance. Eh bien, le peuple de Camargue espère que ses traditions perdureront, malgré les attaques des « anti-tout

pas empêcher les avancées sur d'autres thématiques. Si des avenants ont été signés pour débloquer des crédits en 2021 et 2022, ils ne portaient évidemment que sur des projets inscrits dans les CPER 2015-2020.

Les régions sont prêtes à travailler et signer ces volets mobilité, mais elles n'ont aucune indication sur le calendrier prévu par l'État.

des mandats qui permettront d'engager très concrètement la négociation des volets mobilité pour la période 2023-2027 avec chacune des régions. L'objectif que nous allons nous fixer,

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la mission d'information sur le thème : « Gestion durable de l'eau : l'urgence d'agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement. membres de la mission d'information sur le thème : « Le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique. » En application de l'article 8 de notre règlement, la liste des candidats présentés par les groupes a été publiée. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la désignation des trente-sept membres des commissions spéciales sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, et l'extension du risque incendie, et sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires. En application de l'article 8 , alinéa 3, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes politiques ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

des ratios de soignants par patient. Il n'y a pas que la France qui, soumise à des contraintes budgétaires, a voulu résoudre celles-ci en réduisant le nombre de soignants au lit des malades dans ses hôpitaux. Conjuguée à la stagnation des rémunérations- stagnation qui, les années passant, s'est transformée en baisse -, cette ligne politique visait à contenir les budgets des hôpitaux en actionnant la contrainte du premier poste de dépense, la masse salariale. L'effet fut le même partout : les soignants, mal payés et surchargés de travail, ont commencé à quitter l'hôpital. Si nous voulons rendre à l'hôpital public son attractivité, nous devons répondre à deux problématiques principales celle des rémunérations, en prenant en compte le travail de nuit et le week-end, et celle de la charge de travail, élément fondamental de la qualité de vie au travail pour les soignants, et de la qualité et de la sécurité des soins pour les malades.

Mais la question des rémunérations ne peut à elle seule maintenir ou ramener à l'hôpital des soignants fatigués, lassés de la dégradation des conditions d'exercice de leur mission. Ces soignants, nous les avons longuement écoutés dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête sur la situation de l'hôpital et le

est si précieux dès lors que l'on ne veut pas résumer le soin à des actes techniques, mais respecter en lui les dimensions relationnelle et humaine. L'unanimité de ce constat était frappante et nous nous devons d'y apporter une réponse.

Il faut inverser cette évolution qui sape les fondements des métiers du soin en portant atteinte à leurs valeurs. Il faut revenir à un nombre de soignants par patient plus élevé.

Un effet positif en termes de dépenses est même relevé à moyen terme, car l'augmentation des effectifs est plus que compensée par les coûts évités grâce à la diminution du nombre de complications

Les budgets de tous les hôpitaux, les projets de restructuration de tous les hôpitaux, intègrent des ratios de douze à quinze patients par infirmière quand la moyenne des pays comparables est plutôt de six à En réalité, tout le monde édicte des ratios, mais le législateur, lui, devrait rester silencieux quand ceux-ci sont devenus un puissant facteur de démotivation des soignants, car fondés sur des critères financiers, car déconnectés de la qualité des soins Les travaux préparatoires à notre délibération, et en particulier les nombreuses auditions menées par la rapporteure Laurence Rossignol, que je remercie et dont je salue l'important travail, ont révélé l'unanimité des organisations professionnelles et des syndicats de soignants Des infirmières aux kinésithérapeutes, des sages-femmes aux médecins, tous demandent l'adoption de ce dispositif et le présentent même souvent comme indispensable pour stopper le départ des soignants de l'hôpital. Je veux croire que notre assemblée saura répondre à cette demande. Et d'autant plus largement que le texte adopté par la commission des affaires sociales a intégré les remarques constructives d'un certain nombre d'acteurs sur la nécessaire progressivité des ratios et sur leur adaptation aux spécificités des établissements et des spécialités. Karl Popper, en son temps, a théorisé la nécessité que nous affrontons d'une formule : il faut une règle du jeu et il faut du jeu dans la règle. Nous ne devons abandonner aucun des termes de cette juste position. La souplesse, oui ; le renoncement, non. Aucun motif technocratique ne peut justifier le refus de ratios conformes aux enjeux de qualité et de sécurité des soins quand ceux qui les refusent appliquent sans état d'âme des ratios financiers insupportables pour les soignants. Mes chers collègues, des lits- beaucoup de lits -sont aujourd'hui fermés faute de soignants. Une enquête de l'agence pour l'emploi des soignants menée en 2022 auprès des intérimaires montre que les critères principaux amenant à la décision de quitter l'hôpital et qui pourraient amener à y retourner concernent non pas la rémunération, mais l'adaptation des plannings et un ratio infirmier/patient cohérent. Dans son rapport du 17 novembre 2022- il est donc tout récent -sur les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé, le collège de la Haute Autorité de santé (HAS) confirme que le lien entre les ratios de personnel, la qualité et la sécurité des soins est étayé par la littérature. Alors, mes chers collègues, je sais l'engagement de chacun et de chacune dans notre assemblée pour que nos hôpitaux de proximité, les centres hospitaliers, universitaires non, de nos territoires retrouvent leur attractivité et répondent au mieux aux besoins de santé de nos populations. La mesure que je vous propose aujourd'hui, que la commission des affaires sociales vous propose aujourd'hui, est un élément de réponse fondamental attendu par les soignants. Le Sénat, en adoptant ce texte, enverra deux signaux majeurs. Un premier signal aux soignants, pour leur dire que nous les avons écoutés et entendus et que nous prenons nos responsabilités pour que le sens de leur métier soit respecté, pour que qualité et sécurité des soins soient la règle. Un second signal au Gouvernement, auquel nous demandons de fonder ses décisions à venir sur une véritable approche de santé, non pas en niant la nécessité de choix budgétaires, mais en posant la qualité et la sécurité des soins en déterminant de ces choix. est non plus aux paroles, mais aux actes. Nous pouvons, nous devons prendre soin de nos hôpitaux et de leurs soignants. Je vous appelle à voter cette proposition de loi. La parole

Les soignants sont épuisés. Épuisés de ne plus pouvoir exercer leur métier dans des conditions décentes ; épuisés de devoir assurer des gardes de nuit et de week-end plus nombreuses faute d'effectifs en nombre suffisant épuisés de voir les équipes se déliter, constatant le départ de ceux qui renoncent et le recrutement d'intérimaires qui fragilise encore plus leurs services. Le Ségur, bien que nécessaire, n'a pas répondu à l'ensemble des enjeux.

C'est cette recommandation que Bernard Jomier, qui présidait cette fameuse commission d'enquête, a entendu traduire par la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui. Son principe est simple : établir un nombre minimal de soignants par patient hospitalisé. Celui-ci peut être désigné par les termes « standard » ou « référentiel » : nous avons finalement retenu La commission des affaires sociales- je m'en réjouis -a souscrit au dispositif proposé, qu'elle a amendé sur mon initiative. L'intention est claire : la commission entend s'adresser aux soignants et leur garantir une restauration de leur qualité de vie au travail et de leurs conditions d'exercice.

montrent des effets positifs très clairs liés à la mise en oeuvre de ratios de soignants. Amélioration de la durée moyenne de séjour, baisse de la mortalité ou encore des réadmissions : l'instauration de ratios a des effets favorables en matière de santé publique. du reste pas une surprise. La Haute Autorité de santé constatait en décembre une corrélation reconnue par la littérature entre l'effectif médical et le pronostic des patients. Parallèlement, l'instauration de ratios a des effets tout aussi clairs sur la qualité de vie au travail du personnel soignant : augmentation de l'attractivité, baisse des situations d'épuisement ou de burn-out, soit précisément ce à quoi nous voulons oeuvrer. Pour la commission, rétablir l'attractivité et offrir des conditions décentes d'exercice aux soignants sont des conditions nécessaires pour reconstituer les effectifs et renforcer les équipes. Ce sont les conditions indispensables pour faire revenir les soignants qui ont quitté l'hôpital et pour prévenir de nouveaux départs.

estiment que ces ratios sont complexes à définir, et qu'il est préférable de travailler sur la prise en compte de la charge en soins au quotidien, service par service. Lors des auditions, j'ai beaucoup entendu parler de la « magie » de la charge en soins. soins. Pourquoi cela n'a-t-il jamais été fait ? Voilà trente ans que le sujet est soulevé, et on peine encore à se doter d'outils susceptibles de répondre à ce besoin d'évaluation sans créer de charge supplémentaire. Grâce à la présente proposition de loi, ces outils deviendront une priorité et ils seront enfin pas uniformes, ensuite, car nous sommes allés plus loin en commission, en prévoyant également des distinctions selon la spécialisation et la taille de l'établissement. À situation différente, traitement différent

Le texte prévoit ainsi que ces dernières approuvent l'organisation des soins dans un établissement au regard des ratios fixés. Nous prenons donc en compte les situations particulières, et nous laissons aux soignants la latitude nécessaire dans la définition de leur maquette organisationnelle.

Cette progressivité tient à la nécessité d'évaluer finement les besoins, mais aussi, et surtout, d'engager de manière réaliste les recrutements nécessaires. La commission a, en responsabilité, souligné la distinction entre les ratios de sécurité qui existent déjà aujourd'hui et les nouveaux ratios, établis en vue de garantir la qualité des soins et des conditions d'exercice des soignants. Les ratios qui existent aujourd'hui au nom de la sécurité des patients sont prévus par décret et constituent des conditions requises pour le fonctionnement des établissements.

À ratios différents, conséquences différentes : les ratios de qualité n'entraîneront pas de fermetures de lits. Le fonctionnement des services sera assuré pendant une durée déterminée,

Vous le constatez, madame la ministre, mes chers collègues, il n'est donc point question de rigidité. C'est un changement d'approche qui est proposé : sortir des ratios de performances qui ont fragilisé l'hôpital pour bâtir des ratios de qualité. qualité. Je tiens à souligner pour conclure que la commission des affaires sociales n'oublie pas la nécessité de travailler sur d'autres enjeux directement liés à l'attractivité des métiers et aux conditions de travail, notamment le recrutement.

une brique, mais que celle-ci est indispensable. S'engage avec cette proposition de loi ce que je qualifierai de « loi de programmation », c'est-à-dire une loi qui voit plus loin et qui doit déterminer les moyens à venir. J'espère que notre assemblée adoptera ce texte à la large majorité qu'il mérite, et je souhaite que l'Assemblée nationale et le Gouvernement poursuivent ensuite le travail sérieux engagé par le Sénat.

hémicycle. Face aux tensions auxquelles sont confrontés certains de nos services hospitaliers, en tant que responsables politiques, nous partageons un même sens du devoir. Ce devoir consiste, selon les termes de l'exposé des motifs du texte proposé par le sénateur Jomier, que je remercie d'ouvrir ce débat, « offrir un cadre de travail décent et bientraitant aux professionnels de santé » et à « permettre une prise en charge des patients conforme aux exigences de qualité et de sécurité des soins La proposition de loi dont nous débattons a pour objet d'instituer pour chaque spécialité et type d'activité de soins un ratio minimal de soignants par lit. Plus précisément, de fixer et de faire établir sur le plan national par la Haute Autorité de santé un nombre minimal obligatoire d'infirmiers et d'aides-soignants de jour et de nuit présents au chevet des patients. Si l'intention qui a présidé à l'élaboration de ce texte est tout à fait légitime, son adoption risquerait de nuire à l'objectif fixé, et finalement d'affaiblir la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Lors de son discours de voeux aux acteurs de la santé, le Président de la République a réaffirmé avec conviction que notre méthode pour parvenir à redonner du sens et de l'efficacité au travail des soignants soignants et pour combattre les effets de l'érosion de la démographie médicale consiste à travailler à de meilleures organisations collectives pour favoriser la cohésion de la communauté hospitalière.

Notre objectif est ainsi d'établir un modèle dans lequel les solutions se construisent localement à partir de la charge en soins constatée et des leviers disponibles pour y répondre. C'est pour cela qu'avec François Braun, nous insistons sur la place du service, qu'il faut conforter et renforcer au coeur de l'hôpital. C'est bien cet échelon qu'il convient d'investir pour réinsuffler de la souplesse et retrouver de la pertinence dans des organisations du temps de travail construites avec les soignants. L'établissement de ratios fixes sur une base nationale par la Haute Autorité de santé est à l'opposé de cette méthode. Même en raisonnant par spécialité, même en raisonnant par type d'activité, les besoins de chaque service ne seront jamais les mêmes au même moment,

J'insiste sur ce terme « ressources », qui prend naturellement en compte le nombre des soignants, mais aussi leurs compétences et leur expertise. Il ne s'agit pas de résoudre une équation.

mais en nous appuyant sur une évaluation au cas par cas de la charge en soins et du niveau de ressources adapté à cette charge en soins. Cela suppose aussi de laisser les ajustements spécifiques à la main de ceux qui connaissent le mieux les besoins et les capacités de leurs équipes à y répondre. Le binôme chef de service-cadre de santé est à ce titre fondamental. Il nous faut le soutenir. Avec le ministre de la santé et de la prévention, nous voulons réaffirmer la confiance que nous avons dans ce binôme managérial dans le cadre de la transformation de l'hôpital que nous menons. de santé puissent pleinement se saisir de leur mission de garants de la qualité des soins et de la stabilité des collectifs de leur service. Nous pensons que les managers doivent non pas organiser des cadences et un travail à flux tendu, mais bâtir de nouveaux modèles de développement plus souples, plus adaptés aux contraintes et plus participatifs. Cette confiance, cette marge d'action et cette liberté d'organisation sont essentielles pour que chacun se sente mieux reconnu et valorisé dans son travail. Nous savons qu'un soignant qui se sent bien est un soignant qui soigne mieux. C'est aussi un enjeu important de fidélisation des professionnels, pour que les carrières à l'hôpital public retrouvent des perspectives et toute leur attractivité. C'est de cette manière que nous agirons réellement pour satisfaire à cette double exigence de réponse locale aux besoins des patients et de garanties quant à la qualité de vie des soignants. Il ne s'agit pas de trouver des chemins détournés pour ignorer ou éviter de traiter les problèmes. Oui, certains services sont confrontés à une situation d'insuffisance chronique de personnel. Oui, le manque de soignants est une réalité dans certains services et dans certains modes d'exercice, pour le travail de nuit notamment. Nous devons prendre le sujet à bras-le-corps avec pragmatisme. Nous avons le devoir de trouver les moyens d'y faire face, à très court terme. Toutefois, même si des ratios étaient mis en place avec les meilleures intentions du monde, la question ne se réglerait pas en les « décrétant » dans la loi. François Braun et moi-même restons fidèles à nos convictions : la coercition n'est pas un mode de résolution des problèmes dans les territoires. Dans la mise en adéquation des effectifs avec la réalité des besoins, nous en appelons également à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire à la responsabilisation des directions, qui doivent donner des outils adaptés aux équipes, et à la responsabilisation des équipes de terrain pour se saisir de ces outils. Je parlais de combattre les effets de la diminution de la démographie médicale et des difficultés d'attractivité des métiers de la santé. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés à très court terme, car c'est l'urgence. C'est un travail que nous menons parallèlement et de manière complémentaire aux efforts structurels que nous avons engagés pour nous attaquer aux causes de l'érosion de la ressource soignante et augmenter durablement le nombre des professionnels de santé. nous l'avons rappelé lors de nos voeux aux forces vives, lundi -est de former plus de soignants et de les former mieux. Je pense bien sûr à la suppression du pour les médecins. Je pense au travail que nous menons avec les régions pour remplir des objectifs quantitatifs et qualitatifs de formation de nouveaux infirmiers et infirmières au sein de cursus rénovés et sécurisés.

la mobilisation dans les territoires des leviers locaux d'attractivité afin de faciliter la vie quotidienne de nos soignants, qu'il s'agisse de leur logement, de leur transport, de leur stationnement ou de la garde de leurs enfants. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le constatez, notre politique est globale. Elle est à la croisée des nécessités urgentes et des chantiers de plus long terme. Elle nous permet à la fois de rénover le mode de fonctionnement de nos services hospitaliers à court terme et de travailler à sécuriser leurs effectifs sur le long terme.

En effet, une fois les ratios établis, plusieurs questions très concrètes émergeraient d'emblée. Que se passe-t-il, par exemple, si l'hôpital n'arrive pas à recruter suffisamment pour respecter les ratios imposés par la loi ? Je l'affirme : établir des ratios conduira inévitablement à des réorganisations de l'offre de soins, avec des effets collatéraux nécessitant des rappels de personnel, des fermetures de lits et, dans les cas les plus difficiles, des fermetures de services. Mesdames, messieurs les sénateurs, en tant qu'élus de terrain, vous avez pleine conscience de ces réalités locales. Vous êtes nombreux à nous alerter, à nous écrire, à nous interpeller sur la situation de certains services de proximité dans vos territoires. Si la plupart des services ont tenu face aux tensions de notre système de santé cet été comme cet hiver, c'est parce que les soignants se sont mobilisés avec le soutien des ARS pour y faire face et adapter leur fonctionnement. Ils ont su trouver des solutions managériales pour reconfigurer leurs organisations, travailler avec la médecine de ville pour désengorger les hôpitaux et mobiliser le territoire en appui au fonctionnement des établissements. Si des ratios rigides avaient été en place, de nombreux hôpitaux locaux et services de proximité seraient aujourd'hui fermés, avec des conséquences très dures en termes de prise en charge. Il y a déjà des fermetures ! À l'instar des Assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, les chantiers que nous avons ouverts, et que j'ai mentionnés, doivent venir soulager ces tensions, mais c'est dans un cadre managérial ouvert et flexible, basé sur l'évaluation de la charge en soins réelle, que doivent se décliner ces changements et se déployer les nouveaux soignants que nous formons en ce moment même. Ensuite, les ratios posent des questions éthiques et juridiques majeures. Que faire quand un patient se présente et que sa prise en charge n'entre pas dans la fraction soigné/soignant préétablie ? Que se passe-t-il si un hôpital décide de prendre en charge un patient alors qu'il ne respecte pas les ratios inscrits dans la loi ? Notre mission est bien d'assurer la continuité des prises en charge, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Pour cela, il faut pouvoir s'adapter aux situations afin de proposer la solution la plus efficace et la plus sûre aux malades qui doivent être pris en charge. Imposer mécaniquement des ratios fragiliserait la sécurité juridique des établissements. Il faut se rendre compte que c'est la responsabilité de l'hôpital et de sa direction qui serait directement mise en cause pour tout fonctionnement en deçà des mesures fixées par la loi, y compris en cas d'absentéisme imprévu. Enfin, je constate que le dispositif juridique envisagé aujourd'hui ne s'applique qu'aux établissements de santé assurant des missions de service public. Alors que nous nous appliquons par ailleurs à décloisonner notre système de santé, en en imposant la rigidité de ratios à notre hôpital, le texte aggraverait les iniquités et disparités entre public et privé, que nous combattons justement. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, le Gouvernement est défavorable à l'article unique de la proposition de loi que nous examinons. Cette position ne correspond en rien à un renoncement ou à une hésitation à prendre une position de fermeté. Jamais nous ne reculerons devant des mesures nécessaires pour améliorer l'accès aux soins et conforter les effectifs nécessaires aux lits des patients. Cette position est un choix assumé, car nous ne croyons pas à la coercition, à la centralisation et au modèle unique. Cette position n'est pas un refus. Nous nous inscrivons plutôt dans une politique globale, est de tout faire pour redonner confiance à nos professionnels et leur redonner envie de s'engager à l'hôpital. Il s'agit aussi de sécuriser les collectifs de travail en luttant contre l'intérim cannibale. enfin donner les moyens aux acteurs de proximité, à celles et ceux qui soignent au quotidien, de travailler en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes, en leur laissant la marge de manoeuvre nécessaire pour cela. Cette position, c'est celle de la confiance envers les professionnels de santé, une confiance, je le répète, qui sera accompagnée par le Gouvernement, dans le cadre de la réforme hospitalière et de l'effort inédit de formation que nous menons. Cette position, c'est aussi de vous dire : le travail est pleinement engagé ! Cette proposition de loi est légitime dans ses objectifs. Il nous faut oeuvrer ensemble à une meilleure évaluation des charges de travail de nos soignants, à redonner du temps aux professionnels de santé, pour que nos précieuses ressources humaines soient en adéquation avec les besoins des patients au service de la santé de la population. Associons nos communautés soignantes ; faisons confiance au terrain, en sa capacité à trouver et à coconstruire des solutions. La parole

je comprends aussi parfaitement pourquoi elle est discutée dans cet hémicycle. Notre présidente, Catherine Deroche, l'a rappelé en commission : ce texte résulte

Pour ce qui me concerne, ce sera un « oui, mais ». Oui, car la crise de la covid-19 a été éreintante pour nos soignants, et nombre d'entre eux ont été surmenés. Si cette proposition de loi va dans le bon sens, elle s'inscrit dans un climat toujours aussi tendu dans la communauté Aujourd'hui, en cas de survenue d'un accident médical, par exemple du fait d'un manque de personnel, avec une demande de dommages et intérêts du patient, le juge pourra retenir la responsabilité de l'établissement de santé s'il estime que le nombre d'infirmiers présents n'était pas adapté aux contraintes de service et que ce défaut d'organisation a été à l'origine d'un préjudice pour le patient. Il est donc nécessaire de réformer et d'anticiper. Cette proposition de loi se base notamment sur des expériences étrangères menées en Australie, en Californie, avec des résultats parfois significatifs sur la qualité des soins et le bien-être au travail du personnel soignant.

seulement quelques mois, ne serait-ce qu'en raison du temps nécessaire au recrutement, à la formation et au financement des postes. Si cette proposition de loi laisse jusqu'au 31 décembre 2024 à la Haute Autorité de santé pour définir ces ratios en vue d'une application réglementaire à compter du 1 janvier 2027, il ne faut pas se tromper sur la nécessité d'une réforme dans le système hospitalier. L'attractivité, la rémunération, le bien-être sont des sujets à travailler en profondeur, car ils sont aujourd'hui le coeur d'un système de santé qui s'essouffle. Aujourd'hui, selon plusieurs organisations, près de 10 % des emplois infirmiers ne sont pas pourvus. L'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé suffira-t-elle à résoudre à court terme la pénurie de personnel ? Je n'en suis pas sûr du tout. J'en

Plus largement, mes chers collègues, je veux vous faire partager quelques interrogations. Je ne pense pas que le remède aux maux de notre système de santé réside dans la multiplicité des initiatives législatives ou parlementaires. Je vous ai déjà fait part de cette réflexion lors du débat sur le projet de loi de financement

mais c'est rarement le remède à la pénurie. En vérité, notre système de santé, autrefois une fierté française, est aujourd'hui en grande souffrance et dans une extrême fragilité. Je crois beaucoup plus à une grande loi Santé qui remettrait tout à plat et viendrait redonner du sens au travail Le sens du travail est d'ailleurs une question clé pour la société française d'aujourd'hui, y compris sur la question des retraites. Enfin, il y a un grand risque à mettre le doigt dans l'engrenage de la société de ratios. Des ratios pour les soignants ; demain, des ratios pour les enseignants,

cette proposition de loi vise à établir des ratios de patients par soignant dans les hôpitaux publics et les établissements privés à but non lucratif. Elle entend ainsi apporter une réponse aux difficultés de l'hôpital en instaurant, d'une part, une base légale claire aux ratios de sécurité déjà existants dans certains services- réanimation, soins continus -, et en créant, d'autre part, des ratios dits « qualitatifs », décrits par notre rapporteure, Laurence Rossignol, comme des fourchettes cibles à atteindre en fonction des contextes locaux. Mes chers collègues, l'hôpital va mal ! Les soignants le quittent et des lits ferment. On ne compte plus les exemples de patients restés vingt-quatre, quarante-huit heures sur des brancards dans les couloirs des urgences ; on ne compte plus les témoignages de patients qui ont parfois le sentiment d'avoir été maltraités. Oui, le système actuel est maltraitant, pour les patients comme pour les soignants, alors que l'humain est au coeur de leur vocation. Et il doit revenir au coeur de leur pratique

les soignants doivent, eux, gérer de plus en plus de patients en étant de moins en moins nombreux, ce qui aboutit à une perte de sens, des arrêts maladie et des démissions en pagaille. Les soignants réclament avant tout une amélioration de leurs conditions de travail, et notamment plus de temps consacré au patient.

La rapporteure a évoqué un délai de trois jours pour alerter l'agence régionale de santé en cas d'incapacité à satisfaire les ratios qualitatifs. Trois jours, et ensuite ? L'ARS devra-t-elle aider l'établissement à trouver une solution ou devra-t-elle lui imposer de fermer des lits ? Comment l'ARS pourrait-elle trouver des soignants quand les responsables de l'établissement n'y parviennent pas ? Les hôpitaux ne seront-ils pas tentés de recourir davantage à l'intérim, alors que nous tentons, vainement pour l'heure, de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques ? Malheureusement, les soignants n'apparaîtront pas d'un coup de baguette magique. Aujourd'hui, les établissements veulent recruter, mais il n'y a pas de candidats. C'est pourquoi nous devons former davantage de personnes et, en même temps, améliorer l'attractivité des métiers. C'est un chantier urgent, à mener notamment avec les régions, pour augmenter le nombre de places de formation dans les Ifsi, redonner du sens au métier, réfléchir sur la validation des acquis de l'expérience, développer la voie de l'alternance, qui est encore insuffisamment utilisée, et revoir le financement des formations dans le cadre d'un parcours professionnel. Ensuite, améliorer la qualité de vie au travail, c'est aussi revoir le financement et l'organisation des hôpitaux. Si le Ségur de la santé n'a pas été le déclencheur espéré, il y a urgence à réformer la tarification à l'activité (T2A) et à sortir des indicateurs comme la réduction de la durée moyenne de séjour, par exemple.

de loi risque d'être incantatoire. J'entends l'importance d'envoyer un signal positif aux soignants, mais je crois encore plus à la nécessité d'être efficace. On ne peut plus vendre du rêve aux patients et aux soignants. Vous l'aurez compris, si nous partageons l'intention louable de ce texte, une partie du groupe RDSE reste sceptique sur ses effets réels. Aussi, une bonne partie de ses membres s'abstiendra.

La proportionnalité des moyens hospitaliers était déjà au centre des préoccupations, compte tenu de l'évolution des défis de la santé et du système de soins. Parmi les préconisations formulées, l'amélioration des capacités d'accueil des services d'urgence devait retenir toute notre attention. Aujourd'hui, la conversion d'une de ces recommandations en proposition de loi nous oblige. Le taux d'encadrement des patients, la définition de standards capacitaires et l'utilisation d'indicateurs fiables pour soutenir nos hôpitaux doivent être renforcés. En premier lieu, ces avancées conditionnent un meilleur pilotage de nos politiques de santé. Il s'agit d'un impératif pour préciser les besoins des hôpitaux et pouvoir leur affecter les moyens les plus utiles. Les derniers textes financiers et budgétaires ont notamment permis de préserver les budgets hospitaliers de toute économie malvenue. Une rallonge de 1,1 milliard d'euros a également été décidée pour soutenir les hôpitaux. Afin de permettre une bonne exécution budgétaire et une pleine efficacité de nos politiques de santé, il est nécessaire de disposer d'indicateurs fiables, que la présente proposition de loi contribue utilement à déterminer. En deuxième lieu, il importe que la situation et les seuils concernant l'activité hospitalière se traduisent par des objectifs réalistes. Je veux insister sur ce point, car il a fait l'objet de la plus grande attention et du meilleur engagement du groupe Les Républicains en commission. D'une part, la fixation de ratios minimaux, notamment entre le nombre de soignants et le nombre de lits ouverts, exprime concrètement le souci d'un accueil rationalisé des patients jusque dans les services d'urgence. Un tel ratio doit inclure les personnels de santé effectivement disponibles pour les patients, des infirmiers jusqu'aux aides-soignants. D'autre part, ces ratios doivent être encore

C'est la raison pour laquelle les ratios feront l'objet d'une double adaptation. Ils pourront tout d'abord être modulés pour tenir compte des circonstances locales liées à la population, aux effectifs des hôpitaux et aux moyens disponibles. Ils seront, plus encore, lissés sur les années à venir, selon une politique de santé réaliste, soucieuse d'accompagner ensemble les patients, les soignants et les établissements. Les amendements adoptés en commissions doivent être à cet égard salués. En dernier lieu, ces ratios constituent plus que des conditions d'application de notre politique de santé et de renforcement de nos établissements hospitaliers. Ils portent également une forte charge symbolique pour nos soignants, nos chefs de service et d'établissement. Ils apportent la première pierre au soutien de nos hôpitaux. Les professionnels de santé, nous en avons conscience, sont mus par une vocation à accomplir un service public qui ne doit pas être synonyme de sacrifice permanent pour ceux qui l'assument au quotidien.

qui ne s'accompagnera en pratique d'aucun affaiblissement du service hospitalier et d'aucune fermeture de lits, comme notre collègue rapporteure, Laurence Rossignol, l'a déjà démontré.

Ces difficultés étaient déjà bien présentes avant la crise : manque de personnel, rappel pendant les jours de repos, épuisement. La crise de la covid-19 n'a fait qu'aggraver ces problèmes et beaucoup de soignants ont ainsi choisi de quitter leur profession pour changer de voie. Ces départs dégradent encore davantage les conditions de travail de ceux qui restent, faisant courir le risque de départs en cascade. Le Ségur de la santé a permis de revaloriser leurs rémunérations- il était important de le faire -, mais cela n'a malheureusement pas suffi à endiguer les départs ni à augmenter le nombre de soignants présents auprès des patients. Parfois, les postes financés ne sont pas pourvus. Cette proposition de loi vise à établir et à garantir un ratio minimal de soignants par nombre de lits ouverts dans les services hospitaliers les activités ambulatoires, afin d'assurer aux patients une prise en charge de qualité et de bonnes conditions de travail aux soignants. Aujourd'hui, de tels ratios existent, mais seulement pour certains services- réanimation, néonatologie, soins intensifs, etc.

eux. Prendre soin, ce n'est pas seulement faire des soins, c'est aussi considérer le patient comme une personne qui doit être écoutée et informée. Pour les infirmiers et infirmières, il s'agit de ne pas réaliser les soins au pas de course, d'avoir le temps nécessaire pour observer dans la journée l'évolution de l'état général du patient en fonction de sa pathologie. Les soignants aiment leur métier. Ils prodiguent des soins, mais aussi de l'écoute et de la bienveillance. Or ils sont souvent découragés par l'impossibilité d'effectuer correctement leur travail à cause d'une charge trop lourde et

Bien sûr, le terme « ratio » peut faire peur, car il fait penser à des règles uniformes, strictes, qui ne tiennent pas compte de la réalité propre à chaque établissement. Cette proposition de loi ne doit certainement pas conduire à fermer des lits ni des

devenus très dépendants, une situation qui va s'aggraver nettement d'ici à 2030. Nous attendons donc avec impatience la mise en oeuvre du plan Grand Âge, avec les 50 000 emplois supplémentaires annoncés par le Président de la République, ce qui ferait passer le taux d'encadrement des soignants

nous sommes favorables à cette proposition de loi, qui a pour but d'éviter l'épuisement et le découragement du personnel, d'améliorer la prise en charge globale des patients par plus d'écoute et de surveillance, et ainsi de rendre de nouveau attractif ce très beau métier de soignant. La

nous les avons applaudis depuis nos fenêtres ! Après des années de rationnement, les soignants exigent une perspective de sortie de la crise traversée par l'hôpital public. Le spectre de la dégradation des conditions de travail est vaste : heures supplémentaires subies, travail morcelé, pressé, compressé, vétusté des équipements, ballottement de service en service afin de pallier le manque de personnel. À rebours d'une situation qui empire, cette proposition de loi se veut aussi un signal envoyé aux soignants. Elle ouvre une fenêtre sur un horizon attendu d'effectifs suffisants dans chaque service. Les ratios de soignants permettent d'améliorer tant la sécurité et la qualité des soins que la qualité de vie au travail. Ils sont une partie de la solution. Ils empêchent de faire des effectifs la variable d'ajustement des contraintes budgétaires et limitent les changements incessants d'affectation des professionnels qui gaspillent leur spécialisation, défont les collectifs et produisent souffrance et perte de sens. Dans une lettre ouverte datant de 2022, le collège de la Haute Autorité de santé a souligné « l'importance d'équipes stables partageant une culture commune de qualité et de sécurité des soins Pour autant, les résultats positifs imputés aux ratios, études internationales à l'appui, sont toujours corrélés, donc subordonnés à l'augmentation des effectifs soignants. Le présent texte prévoit un mécanisme d'alerte en cas de constatation d'une incapacité à respecter les ratios qualitatifs au-delà d'une durée de trois jours. Que se passera-t-il ensuite ? Qui aura la responsabilité de sortir de l'injonction paradoxale ?

La distinction introduite entre « ratios de qualité » et « ratios de sécurité » démontre la difficulté de l'équation et de son application. La sécurité des patients et la qualité des soins sont imbriquées, et, en l'état du système de santé, les garanties devraient relever d'une grande loi. Les fédérations hospitalières craignent qu'une équation impossible de plus ne soit imposée au secteur public et au secteur privé non lucratif. En l'état, la crainte de fermetures de lits ou de services n'est pas à négliger, d'autant que l'absentéisme se stabilise à un niveau plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Par conséquent, si nous soutenons l'instauration de ratios dans le secteur sanitaire et appelons à son extension dans le champ médico-social,

l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé, le groupe écologiste votera cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comment ne pas partager le souhait de réduire la charge des personnels soignants, que l'on sait épuisés, ces derniers à rester dans nos hôpitaux ou de faire revenir ceux qui les ont quittés ? Le texte qui nous est soumis vise aussi à assurer une prise en charge de qualité à nos concitoyens grâce à à un encadrement adéquat. Nous partageons ce but, mais est-ce le meilleur chemin ? Présenté comme souple, il risque plutôt de rigidifier l'organisation au sein des hôpitaux, là où, justement, nous nous efforçons de créer de l'agilité pour aller au plus proche des besoins territoriaux. Des ratios de sécurité existent déjà pour certains services, mais, faute des conditions prévues, les capacités d'accueil sont suspendues ou réduites. Ces principes seraient actés dans la loi, alors qu'ils sont, jusqu'à présent, d'ordre réglementaire. Le président du Sénat parlait il y a peu de « sobriété législative dans la loi une mesure qui relève bien davantage du décret ? Le texte propose de créer d'autres ratios, dits « de qualité », sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé. Une révision aurait lieu tous les cinq ans. Le non-respect des ratios qualitatifs au-delà de trois jours serait signalé à l'ARS. Que ferait-on, alors ? Quelles seraient les responsabilités pour les établissements ne parvenant pas à atteindre ces ratios ? L'insécurité juridique d'un tel dispositif et les risques pour la pérennité des services sont à noter. Censé devenir une loi de programmation, ce texte serait appliqué en deux temps. N'est-ce pas faire peser une inquiétude sur les acteurs à court terme ? Alors, oui, je l'ai dit, nous partageons tous la volonté de proposer des solutions aux soignants, mais ce qu'ils souhaitent, à mon sens, ce sont des engagements concrets plutôt que des rigidités à long terme. Je pense aux revalorisations du Ségur, aux mesures de compensation de la pénibilité, notamment pour le travail de nuit,

Je crains que ces ratios ne soient pas la réponse adéquate au regard de l'ampleur de la tâche. Ce texte, dont les intentions sont certes louables, ne peut donc pas, en tout état de cause, représenter une réponse globale aux défis à relever.

Le constat, nous le connaissons et nous le partageons : fermetures de services, annulations d'opérations programmées, démissions dans le personnel soignant, etc. L'hôpital public et ses effectifs sont depuis des années en souffrance et, je dirai même, en détresse. Les périodes de crise et de tensions dans les services hospitaliers se succèdent, et le Ségur de la santé, qui a certes permis une revalorisation salariale, apparaît comme une réponse insuffisante face à l'ampleur des difficultés que rencontre l'hôpital. En effet, plus encore que le trop faible niveau de rémunération, ce sont les conditions de travail dégradées et le manque de temps médical auprès des patients- que dénoncent les soignants -qui entraînent le départ des professionnels. Ainsi, près de 10 % des postes d'infirmière ne sont pas pourvus à l'heure actuelle. Et pour cause ! Ce sont à l'heure actuelle les contraintes budgétaires et non les besoins en soins qui déterminent le nombre d'infirmières dans les services et la composition de l'équipe de soins. Pourtant, nous le savons, le savons, les infirmiers et les aides-soignants jouent un rôle essentiel dans la qualité des soins. Les études scientifiques le montrent : la mortalité des patients augmente dès qu'une infirmière doit s'occuper de plus de six patients. dans nos hôpitaux, une infirmière est, dans la plupart des services, chargée de quinze patients en journée et de vingt-quatre la nuit ! Il paraît donc indispensable de repenser l'organisation du travail à l'hôpital, de changer le paradigme de l'Ondam et de garantir un nombre suffisant de professionnels de santé par patient. Tel est l'objet du texte que nous présentons : assurer à la fois une prise en charge de qualité pour les patients et de bonnes conditions de vie au travail pour les soignants.

médecins, etc. -, d'autre part, les interrogations des directions hospitalières. Cela a amené notre rapporteure à modifier l'article unique en précisant les modalités et le calendrier de l'entrée en vigueur

ont été réalisées en Australie et aux États-Unis. Elles ont montré qu'il existait un lien certain entre l'augmentation de la dotation en infirmières et la diminution de la durée du séjour, des réadmissions, de la morbidité, des erreurs médicales, et, même, des démissions dans le personnel infirmier. Oui, cette mesure sera coûteuse et nécessitera un fort investissement de l'État, mais les études scientifiques le montrent : à moyen et long termes, augmenter les effectifs du personnel soignant constitue un investissement positif sur le plan financier.

dans des services très spécifiques tels que le bloc opératoire, la réanimation et la dialyse. Instaurer des ratios pour chaque spécialité et activité de soins permettrait une amélioration des conditions de travail et contribuerait à rendre les métiers un peu plus attractifs pour les personnels. Ce serait également la garantie d'une meilleure prise en charge des patients. La politique de réduction des dépenses de santé et de non-recrutement de personnel hospitalier a mécaniquement entraîné une augmentation du nombre de patients sous la responsabilité On le sait, l'une des causes majeures des difficultés de recrutement et de la fuite de personnels soignants, en particulier infirmiers, est, plus encore que la faiblesse des salaires, l'augmentation de la charge de travail due au manque d'effectifs. Cette question est d'autant plus importante qu'une étude, parue dans la revue scientifique, a démontré qu'améliorer le ratio soignants par patient diminuait la mortalité, les réadmissions et la durée de séjour. L'idée d'instaurer des quotas est donc fort séduisante. Malheureusement, mes chers collègues, cette proposition de loi ne présente pas que des avantages. En effet, dans le contexte actuel de pénurie, cette proposition risque plutôt de produire des effets pervers. Sans Sans recrutement supplémentaire, et à moyens constants, mettre en place des seuils minimums induit forcément de prendre des effectifs dans tel service pour renforcer tel autre. En d'autres termes, cela revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul Nous avons été alertés par des soignantes et des soignants qui s'inquiètent d'une possible concurrence entre les services pour obtenir des ratios plus importants. Ils craignent, en quelque sorte, de voir s'ouvrir une guerre entre chefs de service. En l'état actuel des choses, ce dispositif peut donc contribuer à accélérer la fermeture de lits, voire à remettre en cause les 35 ces raisons, nous estimons que l'instauration de ratios de soignants par soigné doit aller de pair avec une hausse massive des moyens alloués à l'hôpital. Madame la ministre, vous vous êtes bien gardée de vous engager sur ce terrain. En effet, vous avez fait l'éloge des personnels, affirmé qu'il fallait améliorer les conditions de travail, mais, actuellement, le Gouvernement n'entend pas les revendications des soignants, et n'y répond pas. Dans une tribune parue dans, la sociologue Dominique Méda estimait que la mise en place de tels ratios nécessiterait l'embauche de 100 000 infirmières et infirmiers supplémentaires, pour un coût de 5 milliards d'euros. Madame la ministre, la balle est dans votre camp !

Enfin, nous regrettons le choix de ne pas associer les organisations syndicales à la définition des besoins permettant de fixer, aux côtés de la Haute Autorité de santé et de la commission médicale d'établissement,

personne ne peut ignorer le profond malaise qui touche le monde médical : en témoigne la crise des vocations que ce dernier traverse, celle-là même qui frappe également le corps enseignant. On ne choisit pas cette voie professionnelle par hasard, et c'est heureux ! Il s'agit bien d'une vocation, mais celle-ci ne doit pas devenir un véritable sacerdoce. L'enjeu actuel est de s'assurer que nos hôpitaux puissent disposer de ressources suffisantes afin de garantir une qualité de soins optimale et de bien meilleures conditions de travail aux soignants. En effet, ces dernières années, les hospitalisations conventionnelles ont progressivement été remplacées par des prises en charge ambulatoires. De fait, les patients désormais hospitalisés doivent se voir consacrer plus de temps, car les soins qu'ils demandent sont plus complexes et les pathologies plus lourdes.

Si des ratios sont déjà fixés par décret et sont mentionnés dans le code de la santé publique, notamment en réanimation ou en unités de soins intensifs, dans la plupart des autres services, il n'y a pas de règles en bonne et due forme qui fixent un nombre de soignants par patient. Il convenait de clarifier les choses et de préciser l'articulation des ratios existants, dits de sécurité, avec ces nouveaux ratios de qualité, non moins importants : de cette qualité, évidemment, découle une plus grande sécurité pour les patients. La définition de ces nouveaux ratios serait confiée à la Haute Autorité de santé. Elle les définirait par spécialité et par type d'activité de soin hospitalier, afin de pouvoir répondre le plus précisément possible aux différents besoins. Il était important pour nous de valoriser une approche de terrain aux prises avec les réalités des établissements. Après lecture de la proposition de loi de notre collègue Bernard Jomier,

en commission des affaires sociales- je tiens à remercier tant le travail de sa présidente que celui de Mme le rapporteur -, nous avons garanti aux hôpitaux une capacité d'adaptation en fonction des différentes spécialités et spécificités locales, parfois tout simplement liées à des contraintes architecturales.

revalorisant -que ces métiers deviennent plus attractifs. Sans cela, je le crains, ces emplois resteront non pourvus et ces nouveaux ratios intenables, d'où la progressivité voulue dans la mise en oeuvre de cette proposition de loi. Rappelons que des effectifs suffisants permettent de remplacer plus facilement les absences, ou encore de favoriser la formation en permettant un bien meilleur encadrement des plus jeunes.

à l'approche de la Saint-Valentin, permettez-moi de vous rappeler qu'en politique, comme en amour, il n'y a que les actes qui comptent ! La discussion

La présidente Catherine Deroche l'a rappelé : le professeur Rémi Salomon, président de la CME de l'AP-HP, parle de ce texte comme d'un signal nécessaire à destination des soignants.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans sa version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier. Ce texte n'est pas encore abouti- le rapport de la commission des lois du Sénat ne manque d'ailleurs pas de le relever -, mais il est le fruit d'un travail constructif et transpartisan entre les nombreux groupes politiques de la chambre basse. Je veux d'ailleurs saluer ici les présidentes de groupe Aurore Depuis l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la Cour suprême des États-Unis, six propositions de loi constitutionnelle ont été déposées sur les bureaux des assemblées. Six propositions, six visions différentes, et de beaux débats passés, présents et à venir devant vos deux assemblées. L'importance des initiatives parlementaires dans cette matière démontre que le revirement de jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis a eu l'effet, chez nous, d'un électrochoc.

Disons-le, en la matière, nous ne partons pas de rien et il ne faut pas mésestimer l'oeuvre du Conseil constitutionnel. Celui-ci, depuis sa décision du 27 juin 2001, reconnaît en effet que le droit à l'IVG résulte de « la liberté de la femme qui découle de l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Mais il s'agit à présent d'aller plus loin et de conférer un fondement constitutionnel autonome à l'interruption volontaire de grossesse en l'érigeant explicitement, au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en liberté fondamentale. Pour toutes ces raisons, je persiste et je signe, le Gouvernement soutiendra toutes les initiatives parlementaires qui viseraient à constitutionnaliser le droit à l'IVG. À ceux qui opposent à cette initiative parlementaire que le droit à l'avortement n'est pas menacé en France, je réponds ceci : n'attendons pas qu'il soit trop tard pour le défendre. Le droit des femmes à disposer de leur corps doit être inaliénable. En 1975, Simone Veil expliquait que l'objectif du gouvernement était de créer « une loi réellement applicable, dissuasive, [ ...] protectrice ». Le législateur, au travers de nombreux textes successifs, a atteint ces objectifs. Mais l'objectif que nous visons aujourd'hui est autre. Il s'agit à présent de protéger ce droit en l'élevant au plus haut rang de la hiérarchie des normes, à savoir notre Constitution. Ce faisant, nous donnerions à voir à toutes les femmes - je répète, toutes les femmes -qu'elles ont le choix, que celui-ci leur appartient, et qu'elles sont soutenues par la société tout entière Car, oui, les exemples étrangers partout dans le monde nous le démontrent, une démocratie digne de ce nom ne peut exister sans l'émancipation totale de la moitié de sa population J'appelle votre attention sur la nécessité de ne pas se tromper de débat. J'entends évidemment la commission des lois lorsqu'elle pointe qu'une telle inscription ne résoudrait pas les difficultés concrètes d'accès à l'IVG, qui peuvent se rencontrer sur le terrain.

Si les modalités d'exercice du droit à l'interruption volontaire de grossesse doivent pouvoir continuer à être encadrées par le législateur, car il s'agit du niveau normatif le plus le plus adapté pour le faire, le droit à l'interruption volontaire de grossesse lui-même ne doit pas être entravé, restreint ou, pis, aboli. Une garantie constitutionnelle peut nous l'assurer pour l'avenir. Et ce pour une raison que j'avais évoquée devant vous au mois d'octobre dernier : constitutionnaliser le droit à l'IVG, c'est s'assurer que ceux qui auraient ce néfaste projet ne puissent le faire sans sans l'accord du Sénat. Oui, inscrire le droit à l'IVG dans notre Constitution, c'est garantir que le Sénat aura le dernier mot pour protéger celui-ci, comme il en a en déjà protégé tant d'autres, dans la noble mission qui est la sienne. Vous l'aurez compris, tout comme la commission, le Gouvernement n'a pas changé d'avis : il est, lui, favorable à l'inscription du droit à l'IVG dans notre Constitution. J'en viens maintenant au sujet qui est sans doute le plus complexe, comme en témoignent les nombreuses versions et amendements déposés dans les deux chambres : je veux bien sûr parler de l'emplacement et de la rédaction de cette inscription. Je le dis d'emblée, il nous faut faire montre de la plus grande humilité relativement à ces deux questions. Nul ne détient la vérité révélée et les propositions méritent toutes d'être examinées pour les avantages qu'elles contiennent, aussi bien que pour les réserves qu'elles entraînent. L'emplacement de ce droit au sein de la Constitution n'est pas une question purement symbolique. C'est avant tout une question juridique. je l'ai déjà dit, il ne faut toucher à notre Constitution, selon la formule désormais consacrée, que d'une main tremblante. La commission des lois ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a relevé qu'une telle disposition devait trouver sa place dans notre Constitution, pour s'y fondre, au risque, sinon, de la fragiliser. Le choix de cet emplacement sera également la traduction de la portée que le Parlement a voulu lui assigner. Il participera directement à donner tout son sens à la reconnaissance de ce droit. À cet égard, M. le sénateur Philippe Bas a déposé un amendement ayant pour objet, outre qu'il propose une rédaction alternative, de placer la reconnaissance de ce droit à l'article 34 de la Constitution. Je l'ai dit, cette proposition, comme les précédentes, mérite un examen attentif. Sans déflorer les débats que nous aurons dans quelques instants,

Elle renvoie en effet entièrement au législateur le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les femmes peuvent recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est, très exactement, l'état de notre droit. Vous le savez, il résulte déjà de l'article 34 de la Constitution qu'il revient au seul législateur de prévoir les garanties, tout comme les limites, du droit à l'avortement. C'est ce qu'il a fait encore récemment, par la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement, ce dont, par ailleurs, je me réjouis. J'entends votre argument cet alinéa, en faisant référence à cette liberté qu'il revient à la loi d'organiser, consacrerait implicitement cette liberté au niveau constitutionnel. Le doute subsiste sur la réalité de cet effet. Je comprends et partage par ailleurs votre souci de laisser une certaine marge de manoeuvre au législateur : il est en effet souhaitable que les conditions dans lesquelles le droit à l'avortement s'exerce puissent évoluer avec le temps. L'Assemblée nationale a, quant à elle, retenu la création d'un nouvel article 66-2. Cet emplacement a été choisi par les députés afin de donner une chance

Le sujet reste donc ouvert sur ce point. Par ailleurs se pose bien évidemment la question de la rédaction de cette inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Là encore, et à plus forte raison, il nous faut être humbles face à la tâche. Chaque mot doit bien évidemment être réfléchi, pesé, justifié. Et il ne s'agit pas là d'une entreprise très aisée. Après le refus net du Sénat de constitutionnaliser le droit à la contraception, l'Assemblée nationale a fait un premier pas. Elle a ainsi renoncé, par son vote, à l'inscription du droit à la contraception dans la Constitution, recentrant ainsi la proposition sur la constitutionnalisation de l'IVG. Pour motiver son refus, la commission des lois a, à son tour, relevé, à bon droit, les risques d'une rédaction inaboutie

Il est vrai, comme je l'ai indiqué devant l'Assemblée nationale, qu'une rédaction inadaptée pourrait conduire à consacrer un accès sans aucune condition à l'interruption volontaire de grossesse, par exemple à des IVG réalisées bien au-delà de la limite légale en vigueur. Une écriture mal jaugée pourrait également se révéler trop rigide et empêcher une adaptation possible du dispositif actuel, si celle-ci était nécessaire,

la tâche est ardue, mais la volonté est claire. Le Parlement se mobilise comme jamais auparavant pour consacrer le droit à l'IVG dans la Constitution. Le Gouvernement est venu, devant chaque assemblée, soutenir les initiatives, d'où qu'elles émanent, en participant aux débats, dans le rôle qui est le sien. La navette parlementaire fait son oeuvre, car je crois comprendre que l'Assemblée nationale a pris acte du premier refus du Sénat et vous présente une version prenant en compte un certain nombre de craintes. Comme je vous l'ai dit, toutes les craintes ne sont pas levées, car l'oeuvre est complexe. Mais l'espoir est permis, l'espoir que le Parlement, avec l'appui du Gouvernement, poursuive ses travaux pour trouver un accord. Il y va du droit des femmes à disposer de leur corps. Cela seul devrait suffire à nous convaincre tous.

Notre responsabilité de législateur est d'élaborer une norme avec une certaine hauteur, retenue et maîtrise, quand celle-ci tend à réviser la Constitution. Le 24 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un texte porté par la présidente du groupe La France insoumise (LFI) visant, de nouveau, à inscrire dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, il est soumis à notre examen. à introduire un nouvel article 66-2 au sein du titre VIII consacré à l'autorité judiciaire, article selon lequel « la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse La question n'est donc pas de savoir si nous sommes pour ou contre l'IVG. Ne nous laissons pas enfermer dans une lecture simpliste, binaire et, parfois, manichéenne. La véritable question qui nous est posée est la suivante : faut-il réviser la Constitution pour y inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse ? Faut-il modifier la norme supérieure pour reconnaître la liberté pour toute femme de mettre fin à sa grossesse ? Nous pensons que, même si l'opinion publique est forte, cette idée est une fausse bonne idée. En effet, si les députés ont supprimé la référence à la contraception, cette évolution n'est pas de nature à lever les doutes, déjà émis par le Sénat, sur la pertinence de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Le 19 octobre dernier, notre assemblée a rejeté une proposition de loi similaire présentée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse [ ...] ». La liberté de la femme d'avorter est, aujourd'hui, pleinement protégée par la loi du 17 janvier 1975 portée par Simone Veil, loi qui fait désormais partie intégrante de notre patrimoine juridique, et à laquelle le Sénat s'est toujours montré fortement attaché. L'accès à l'IVG n'a jamais cessé d'être conforté par le législateur : allongements successifs des délais, élargissement des praticiens pratiquant des IVG, amélioration de la prise en charge financière, suppression du critère de « situation de détresse » ou encore du délai de réflexion préalable. Certes, le Conseil constitutionnel n'a jamais consacré de droit constitutionnel à l'avortement, mais il l'a toujours jugé conforme à la Constitution, les quatre fois où il s'est prononcé sur le sujet : en 1975, en 2001, en 2014 et en 2016. Le Conseil constitutionnel, peu importe le contexte ou l'époque, n'a donc jamais remis en question ce droit fondamental des femmes. Depuis sa décision du 27 juin 2001, il rattache le droit à l'IVG au principe général de la liberté de la femme découlant de l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qu'il concilie avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation. La jurisprudence établie du Conseil constitutionnel offre d'ores et déjà une protection forte de cette liberté de la femme. lors, existe-t-il un réel danger de remise en cause de l'IVG en France ? Aucun groupe politique n'a jamais indiqué vouloir remettre en cause ce principe : il n'est donc pas crédible de soutenir que ce droit est menacé en France, de la même manière qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays de l'Union européenne. À cet égard, la situation institutionnelle de la France n'est en rien comparable à celle des États-Unis. Dire le contraire, c'est méconnaître la réalité profonde de la décision de la Cour suprême du 24 juin 2022,, qui a renvoyé aux États fédérés la compétence pour légiférer sur l'avortement. En France, la situation est radicalement différente. Notre République est une et indivisible. Le législateur national dispose ainsi d'une plénitude de compétences et les lois sont les mêmes pour tous. En définitive, le dispositif « anti-Trump » envisagé par cette proposition de révision constitutionnelle n'a pas lieu d'être en France. Je préfère donc rester fidèle aux conclusions rendues par le comité présidé par Simone Veil, en décembre 2008, qui avait recommandé de ne pas modifier le préambule ni d'intégrer dans la Constitution « des dispositions de portée purement symbolique ». Car ce n'est pas un symbole qui résoudra l'accès effectif à l'interruption volontaire de grossesse. Je m'indigne, tout comme vous, des difficultés que rencontrent certaines femmes pour interrompre leur grossesse. Il est profondément inacceptable que des femmes qui souhaitent recourir à l'IVG ne puissent le faire dans de bonnes conditions, en particulier dans certains territoires. Mais est-ce que la constitutionnalisation résoudra ce problème ? Malheureusement non, une telle voie est illusoire. L'accès effectif à l'IVG en France impose des moyens supplémentaires pour le planning familial, impose l'accès à un médecin dans tous les territoires, impose le développement des mesures de prévention auprès des jeunes, impose un ensemble de mesures concrètes, d'ordre réglementaire ou législatif, mais en aucun cas de nature constitutionnelle. Il est clair, par ailleurs, que la Constitution du 4 octobre 1958 n'a jamais été conçue pour qu'y soient intégrées toutes les déclinaisons des droits et libertés énoncés de manière générale dans son préambule. Pourquoi, dès lors, se limiter à l'IVG et ne pas constitutionnaliser d'autres manifestations de la liberté, qui n'ont pas non plus, en tant que telles, valeur constitutionnelle ? Pourquoi ne pas inscrire dans le dur tous les droits et libertés reconnus par le Conseil constitutionnel ? Pourquoi ne pas inscrire demain tous les droits liés à la bioéthique ou à la fin de vie ? Parce que notre Constitution ne doit pas être un catalogue de droits au contenu limité. ce débat sur la constitutionnalisation n'est pas aujourd'hui abouti. La proposition de loi constitutionnelle dont nous débattons, tout comme les multiples initiatives législatives, soulève l'épineuse question de la manière de réviser la Constitution. La difficulté de trouver une place pertinente parmi les dispositions constitutionnelles témoigne de l'absence de cohérence de la proposition de révision avec le texte de la Constitution. Son intégration au sein du titre VIII relatif à l'autorité judiciaire, juste après l'abolition de la peine de mort, a de quoi surprendre. Les propositions d'inscription à l'article 34, qui détermine le domaine de la loi, ou à l'article 1, qualifié d'« âme de la Constitution » par le doyen Carbonnier, ne sont pas plus satisfaisantes.

Or le législateur doit pouvoir en fixer les conditions, comme pour toutes les libertés publiques : l'avortement ne saurait être un droit absolu, sans limites. Enfin, je réitère les mêmes réserves de procédure qu'en octobre dernier : il convient d'avoir un débat serein sur les « mérites » d'une constitutionnalisation de l'IVG. Si ceux-ci étaient réellement démontrés, l'introduction dans la Constitution devrait suivre la voie d'un projet de loi constitutionnelle afin d'éviter de mettre au coeur de l'actualité, par un référendum, un sujet sur lequel il n'y a pas de débat public. Pour toutes ces raisons, étant très attachée au droit à l'interruption volontaire de grossesse, composante de la liberté de la femme, je vous invite à ne pas adopter cette proposition de loi constitutionnelle.

un texte inutile et dangereux visant à constitutionnaliser le droit à l'avortement. Je commencerai par citer un rapport sur l'inflation normative remis la semaine dernière par nos collègues Françoise Gatel et Rémy Pointereau. Même s'il concerne les normes applicables aux collectivités territoriales, leur propos peut tout à fait être élargi à notre sujet.

à son tour. Si tant est que cette révision soit adoptée, qu'aurez-vous changé au quotidien des femmes de France ? Rien ! Pourquoi, alors, s'opposer à ce texte, me direz-vous, mes chers collègues ? Parce que son inutilité modifie l'esprit de la Constitution : l'État de droit se transforme en tas de droits. Dès lors que le pouvoir constituant s'introduit dans la chambre à coucher, les revendications privées prennent le pas sur le bien commun. La cède le pas à la. La République devient la « Réprivée », c'est-à-dire l'anarchie et la fin de la société en refusant de rejeter ce texte de révision, vous multipliez les normes à valeur constitutionnelle contradictoires et renforcez les pouvoirs d'arbitrage des juges, au détriment du Parlement, donc de la démocratie. de la démocratie. Si je me permets de défendre ce point de vue devant vous, c'est avec d'autant plus de vigueur et d'honnêteté que je le fais sans aucun intérêt électoral, mais avec le souci de l'intérêt général. On ne joue pas avec les textes juridiques sans conséquence politique. La loi Veil a dépénalisé l'avortement voilà quarante-huit ans. Vous souhaitez aujourd'hui en travestir l'esprit, en l'établissant comme un objectif de société. Contrairement à ce que vous affirmez, l'avortement n'est pas menacé en France ; ... Il l'est, par vous ! ... ce droit a même été renforcé. Le pays ne s'est pas mis en grève générale, hier, pour l'interdire ! En revanche, la natalité, elle, est réellement menacée

L'ère des conséquences est venue. Sachons tirer les enseignements qui s'imposent avec le sens des responsabilités ! Et de la mesure ! Je vous propose donc, mes chers collègues, de couper court à cette instrumentalisation de la Constitution, en rejetant dès à présent ce texte inconséquent et idéologique présenté, dois-je le rappeler, par La France insoumise.

Aucun pays n'est jamais à l'abri d'une majorité politique porteuse des idées que vous défendez- les Français nous en préservent ... -, susceptible d'abroger les dispositions autorisant l'avortement et la contraception ou d'en restreindre considérablement l'accès.

J'ai une petite divergence avec vous, madame la rapporteure : vous dites que le droit à l'avortement n'est pas menacé dans notre pays. Mais, aux États-Unis, quand il a été permis aux femmes d'avorter, personne ne pouvait imaginer qu'un jour

Le scrutin est ouvert.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte dont nous débattons aujourd'hui a été rejeté en commission mercredi dernier, trois jours après l'organisation d'une manifestation « pour la vie » à Paris. Rien de nouveau sous le soleil sénatorial : un texte similaire avait déjà été rejeté en octobre dernier. Si le recours à l'avortement est protégé en France par la loi Veil du 17 janvier 1975, il ne bénéficie pas pour autant de la protection la plus forte qu'offre notre droit. Sanctuariser, en le faisant entrer dans la Constitution, ce droit fondamental de la femme à disposer de son corps le mettrait à l'abri à l'abri des tempêtes politiques françaises. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans des pays de l'est de l'Europe, comme la Pologne ou la Hongrie, et dans une grande démocratie, démocratie, les États-Unis, sous la pression des conservateurs. L'Italie risque à son tour de s'engager dans cette voie de la régression. Notre collègue Philippe Bas a proposé une nouvelle rédaction de la formule retenue par l'Assemblée nationale, en substituant à la notion de « droit d'accès à l'IVG » celle de « liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse

temps encore devrons-nous nous battre pour une reconnaissance pleine et entière du droit des femmes à disposer de leur corps, à choisir leur maternité ? Les hommes choisissent bien leur paternité et jouissent bien du droit de reconnaître ou non leur enfant ... Pourquoi vouloir toujours,

De surcroît, seul ce véhicule législatif permettrait d'éviter la case du référendum, très périlleuse dans le contexte politique actuel, au cas où les deux chambres se mettraient d'accord sur un texte ; à moins, bien sûr- je ne l'espère pas -, que le but inavoué de l'exécutif soit de faire traîner les choses ou de les rendre difficiles. La parole est

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, chacun a en tête la volte-face historique de la Cour suprême américaine, qui est venue rappeler combien l'accès à l'avortement demeure très inégal et fragile dans le monde.

... Si nous sommes attachés à la défense de l'IVG comme liberté pour les femmes et pour les hommes qui les accompagnent, nous sommes également attachés à notre Constitution comme texte fondamental et précieux. Chacun connaît ici la formule de Montesquieu : on ne touche à la Constitution que d'une main tremblante. De toute évidence, le choix de placer cette disposition dans un chapitre consacré à l'autorité judiciaire ne saurait convenir. L'article 34 aurait paru plus opportun, en tout cas moins inapproprié. J'ai également entendu certains arguments qui ne m'ont pas convaincu : « nous sommes en France et non aux États-Unis », plaident ceux qui nient la tendance mondiale et européenne à une forme de recul des droits et des libertés fondamentales des femmes. Au contraire : si d'autres reculent, soyons fiers de montrer le chemin inverse, le chemin qui refuse la régression ! Par ailleurs, avance-t-on, la constitutionnalisation serait illusoire, parce qu'elle ne résoudrait pas les problèmes d'accès à l'IVG. Évidemment ! Mais à quoi faudrait-il s'attendre ?

Les problèmes d'accès et de réalisation concrète ne sont globalement pas des problèmes constitutionnels : c'est au législateur et au pouvoir réglementaire de les régler. Notre Constitution doit afficher des principes, des valeurs et des objectifs. Elle indique la finalité de notre droit, celle à laquelle il ne saurait déroger. De toute évidence, la garantie donnée à la liberté des femmes d'interrompre leur grossesse trouvera sa place dans un tel corpus. Et il me semble trop précaire de se limiter à la seule interprétation jurisprudentielle du Conseil constitutionnel. Pour reprendre les mots de notre collègue Stéphane Artano, un revirement de jurisprudence et d'interprétation serait trop simple à justifier : on nous expliquerait que l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur lequel le Conseil appuie sa jurisprudence, ne se réfère, au sens strict comme au sens historique, ni à l'IVG ni à la contraception.

permettez-moi tout d'abord de saluer l'extrême pertinence et la vigueur de la présentation du rapport de la commission des lois par Mme Agnès Canayer. Elle justifie amplement notre refus de voter ce texte. Je reprendrai seulement quelques-uns des arguments qu'elle a énoncés, en m'attachant au texte de cette proposition

la rédaction proposée ne définit pas ce qu'est le droit à l'interruption volontaire de grossesse, le présente comme un absolu, une sorte de créance sur la société, et ne prévoit de garanties par le législateur que pour son « effectivité », qui relève plutôt de l'organisation du système de santé, et pour son « égal accès », qui est naturellement une mesure sociale tout à fait estimable, mais qui n'est pas au coeur du débat. Ce qui est au coeur du débat, en revanche, c'est la substance de ce droit indéfini à l'interruption volontaire de grossesse que les auteurs de cette proposition de loi prétendent vouloir reconnaître. Comme M. le garde des sceaux l'a suggéré dans son intervention, l'idée que ce droit serait illimité, le mettant à part de toutes les autres libertés constitutionnelles, n'est pas exclue par la rédaction adoptée Et il nous semble que l'on ne peut reconnaître un droit ou une liberté sans en prévoir aussi les conditions, c'est-à-dire les limites. C'est précisément ce qui fait l'équilibre de la loi Veil jusqu'à l'achèvement d'un certain délai, c'est la liberté de la femme qui prévaut ; après l'achèvement de ce délai, c'est la protection de l'enfant à naître, dont je m'étonne que personne n'ait parlé.

de la République, et l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. On a décidé également que nul ne peut être condamné à la peine de mort. La Constitution est donc bien un lieu qui permet d'accueillir des libertés que le pouvoir constituant, qui est souverain

Cette contre-proposition vise à garantir l'équilibre de la loi Veil : elle reprend l'énoncé d'une liberté qui a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2001 et elle consolide cette liberté. Mais elle prévoit aussi que le législateur en détermine les conditions, donc les limites, comme l'a prévu la loi Veil. est que l'on ne peut pas sortir de cette équation : il n'y a pas de droit absolu ; il y a une liberté déjà reconnue et que nous pouvons écrire dans la Constitution, mais à la condition que soient conciliés les droits de la femme enceinte de mettre fin à sa grossesse et la protection de l'enfant à naître après l'achèvement d'un certain délai. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Monsieur le garde des sceaux, vous avez dit tout à l'heure, rappelant une formule célèbre, qu'il ne fallait toucher à la Constitution que d'une main tremblante. Les vôtres, de mains, sont restées dans vos poches

pour engager un processus qui aurait de meilleures chances d'aboutir. Très bien ! Vous restez sur le banc de touche, libre à vous ! C'est un confort que nous ne voulons pas vous donner durablement, car le verrou du Sénat peut être levé et vous serez alors mis face à vos responsabilités.

Il vise à faire de l'IVG un droit constitutionnel. Sa rédaction était initialement identique à celle du texte rejeté par notre chambre en octobre dernier.

Ce régime, comme bien d'autres, est le fruit d'un équilibre délicat, qui concilie, en l'espèce, la liberté de la mère, d'une part, et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, d'autre part. Certaines évolutions législatives étrangères font craindre un recul des libertés. Un revirement de jurisprudence de la Cour suprême américaine a ainsi rendu aux États fédérés de ce pays le choix d'interdire ou d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse ; il s'agit d'un retour en arrière manifeste.

Les reculs de cette liberté se traduisent par des poursuites pénales, tant pour la mère que pour le médecin. Comme nos concitoyens, ces évolutions nous inquiètent. Dans notre pays, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas, à l'heure actuelle, politiquement

Cependant, ce qui menace l'IVG, c'est bien davantage le manque de moyens et de médecins, qui transforme cette intervention en parcours de la combattante. Le Gouvernement s'est dit favorable à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse.

Dans ces conditions, il sera difficile d'expliquer pourquoi l'Assemblée nationale et le Sénat auront débattu longuement et à plusieurs reprises d'une éventuelle constitutionnalisation sans que ces débats aient en rien amélioré l'accès de nos concitoyennes à l'IVG. Nous l'avons dit, notre groupe est très attaché aux libertés individuelles, notamment à la liberté d'interrompre une grossesse. Nous souhaitons également que nos concitoyennes bénéficient d'avancées concrètes. À cet égard, il nous semble nécessaire de densifier l'offre de soins sur notre territoire.

Trop de femmes sont encore contraintes de se rendre à l'étranger pour avorter. Que ces femmes soient mineures ou non, qu'elles aient été victimes d'agression ou non, l'interruption volontaire de grossesse est toujours une épreuve. Il est de notre devoir d'accompagner au mieux les femmes qui y ont recours. Les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires sont unanimement favorables à la liberté d'avorter. Certains s'interrogent sur l'intérêt de son inscription dans la Constitution. Chacun votera donc selon ses convictions. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas part au vote, car les termes de la loi Veil me paraissent suffisamment équilibrés.

je souhaite d'abord saluer le travail de l'Assemblée nationale- ce vote qui a rendu si fiers les Françaises et les Français -et le sens de l'intérêt général qui a été celui de Mathilde Panot, d'Aurore Bergé et de toutes celles et tous ceux qui, à gauche comme à droite, ont su se rassembler autour d'un impératif bien plus grand que nos désaccords politiques. La loi Veil, que tant d'entre nous ont évoquée ici, et dont il sera encore question au cours du débat, point de départ de l'accès des femmes au droit à l'avortement en France, a nécessité, comme tant d'autres victoires politiques, la réunion de trois éléments. la mobilisation des féministes qui, comme toujours, des années durant et depuis des décennies, ont battu le pavé et mis leur vie en danger pour sauver tant d'autres de l'horreur et pour imposer la reconnaissance de ce dû le plus fondamental, celui que nous avons à disposer de nos corps, à contrôler notre fécondité et, plus largement, à maîtriser nos vies. la détermination et la responsabilité de la gauche, une gauche qui a su, à un moment donné de l'histoire et quand bien même la loi Veil était loin, bien loin, de notre idéal rendre possible l'imparfaite, mais nécessaire victoire. Le troisième élément- et c'est profondément de cela, au fond, dont il est question aujourd'hui -est la dignité d'une certaine partie de la droite qui, en dépit des pressions, du conservatisme et de l'idéologie violemment sexiste et misogyne qui pétrissaient alors une bonne partie de ses rangs, s'est alliée à un combat dont aucun digne représentant de la Nation ne pouvait continuer à freiner l'aboutissement. Nous sommes, aujourd'hui, dans une situation foncièrement similaire. Parce qu'elle est tant attachée à ce qui constitue l'une des conditions les plus fondamentales de l'égal accès à la citoyenneté, la population française, à hauteur de 86 %, souhaite voir le droit à l'IVG entrer dans la Constitution. Parmi ces 86 se trouvent nombre de vos filles, de vos petites-filles et de leurs amis. Ce sont toutes celles et tous ceux qui savent dans leur chair que, quand il s'agit d'IVG, aucune protection n'est superflue et qu'il vaut toujours mieux trembler d'une main pour protéger des droits que se tétaniser pour refuser de le faire. Pas pour le symbole ou l'esthétique, raison de la responsabilité immense conférée par la conscience aiguë que nous avons des menaces qui planent toujours sur les droits des femmes et de la force de ce message d'espérance que la France peut aujourd'hui envoyer au monde entier. Si la France n'est pas un pays magique, protégé de la marche du monde, immunisé contre les reculs, elle est aujourd'hui un pays tout particulier. Un pays que regardent non pas seulement les Américaines, aussi les Polonaises, les Maltaises, les Hongroises, les Allemandes, les Italiennes, les Iraniennes, les Chiliennes. Un pays qui peut, dans cette période si sombre pour les droits des femmes, tracer enfin un chemin d'espoir et de progrès. Je ne sais pas, mes chers collègues,

alors tout le mal du monde à expliquer à leurs petites-filles qu'ils ont tout fait pour ne pas les protéger ! Pour ce qui nous concerne, comme dans tous les moments de bascule de l'histoire, nous saurons toujours où est notre responsabilité. Nous sommes prêtes et prêts à voter un texte qui,

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 19 octobre dernier, le Sénat rejetait la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Mélanie Vogel visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Outre les arguments avancés lors de ces débats, sur lesquels je ne reviendrai pas, nous retiendrons de ce vote le signal malheureux envoyé à nos concitoyens, particulièrement aux femmes. Ne soyons pas sourds à leur demande : ils nous regardent.

Malgré cela, en dépit des solides arguments avancés, nous n'avons pas réussi à obtenir une majorité en octobre dernier pour protéger et garantir le droit à l'interruption volontaire de grossesse, en l'inscrivant dans notre Constitution. Qu'attendons-nous, mes chers collègues ? Ne nous trompons pas de débat : il s'agit bien ici d'empêcher un retour en arrière qui suscite la crainte d'un bon nombre de nos concitoyens. Nous avons de nouveau l'occasion de voter en ce sens, saisissons-la En constitutionnalisant le droit à l'IVG, notre pays ferait oeuvre de pionnier en la matière. Ne sous-estimons pas la puissante portée symbolique d'un tel acte vis-à-vis de l'Occident. Fidèle à sa vocation universaliste, la France enverrait un message fort aux pays où le droit à l'avortement est bafoué ou inexistant. Elle défend vigoureusement sur la scène internationale les droits des femmes ; alors, allons plus loin ! Je tiens à saluer notre collègue Philippe Bas qui, dans un esprit constructif, propose de réécrire l'article unique dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Bien que son amendement prévoie que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse, il ne consacre pas pour autant le droit à l'IVG comme un droit autonome. Pour aller plus loin, mes chers collègues, j'ai déposé un sous-amendement dont l'adoption constituerait, selon moi, une avancée rédactionnelle significative, notamment en faisant apparaître les notions d'effectivité et de libre accès à ce droit.

Contrairement à ce vous affirmez, madame la rapporteur, l'inscription dans notre loi fondamentale d'un droit garanti depuis près de cinquante ans ne semble pas constituer un « changement de nature de la Constitution dommageable ». Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à considérer que la constitutionnalisation du droit à l'IVG serait parfaitement compatible avec notre tradition juridique. C'est pourquoi une large majorité de sénateurs du groupe RDPI soutiendra ce texte,

Rappelons-nous le long chemin parcouru, la lutte âpre et parfois violente que les femmes ont menée pour obtenir, par la première loi Veil du 17 janvier 1975, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. N'oublions pas toutes ces femmes criminalisées pour avoir avorté ou pour avoir aidé d'autres à le faire. N'oublions pas toutes celles qui sont mortes faute d'avoir eu accès à des conditions dignes pour pratiquer un avortement. La constitutionnalisation de l'IVG s'inscrit dans cette longue histoire des luttes des femmes pour leurs droits. Cela a été rappelé, notre Constitution est la règle la plus élevée de l'ordre juridique, elle organise notre vie institutionnelle, mais elle définit aussi les valeurs et principes qui fondent la communauté politique ; elle traduit notre contrat social. le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, « l'égalité de genre impose [ ...] de tenir compte des besoins de santé des femmes, qui diffèrent de ceux des hommes ». Si ce principe avait été connu des rédacteurs du préambule de la Constitution de 1946, son article 3 qui garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes aurait consacré la liberté reproductive spécifique des femmes. La liberté reproductive des femmes est la condition de l'égalité entre les sexes et doit figurer à ce titre dans le texte qui fonde notre communauté. Ce serait notre fierté Ce serait notre fierté et notre honneur que d'être le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution le droit des femmes à disposer de leur corps.

Pourtant, certains pensent qu'il serait inutile de protéger le droit à l'IVG au motif que la législation actuelle le protégerait déjà suffisamment. Mais, comme l'a dit précédemment le garde des sceaux, ne sera-t-il pas alors trop tard pour légiférer si des forces rétrogrades prennent le pouvoir et décident de s'attaquer à ce droit ? N'avez-vous pas vu les manifestations hostiles au droit à l'avortement qui se sont tenues au cours des derniers mois, notamment dans les rues de Paris il y a quelques jours, rassemblant plusieurs milliers de personnes ? D'autres affirment que le droit à l'IVG serait déjà garanti constitutionnellement au titre des libertés fondamentales : cela résulte, selon nous, d'une incompréhension. Si le Conseil constitutionnel n'a pas conclu à une inconstitutionnalité depuis sa décision initiale sur la loi Veil en 1975, puis pour chacune de ses modifications législatives, il n'a cependant jamais formellement reconnu l'IVG comme un droit fondamental. Ces lois ont été validées au motif qu'elles respectaient un équilibre entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article II de la Déclaration de 1789,

Mais pourquoi opposer la constitutionnalisation de l'IVG et la question de son accès ? Ne pourrait-on pas, à la fois, améliorer l'accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire et donner une protection supplémentaire à ce droit, en le constitutionnalisant ?

c'est penser que la France serait une sorte d'îlot protecteur et protégé dans une Europe et un monde qui, concernant l'ensemble des droits

un mot, enfin, sur la proposition de notre collègue Philippe Bas qui s'engage dans cette constitutionnalisation avec une rédaction différente, qu'il nous a détaillée. Cette présente selon nous deux faiblesses. Tout d'abord, elle n'est pas conforme au dispositif retenu à l'Assemblée nationale et ne permet pas à ce stade de vote conforme

par notre collègue a pour vertu de s'engager sur le chemin de la constitutionnalisation. Au fond, rappelons-nous que la première loi Veil n'a pu être adoptée que grâce à un travail

Républicain la soutiendra : elle est positive, même si elle est imparfaite. Monsieur le garde des sceaux, je reprendrai à mon compte les propos de Philippe Bas. Vous avez fait état d'une analyse très fournie et intéressante, mais nous avons envie de vous voir concrétiser cette analyse

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, Gisèle Halimi affirmait déjà en 1973 : « Il y a dans le droit d'avortement de la femme une revendication élémentaire, physique, de liberté. Plusieurs d'entre vous, mes chers collègues, ont dit que ce droit existait et qu'il était reconnu depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, à la suite des mobilisations de femmes, d'associations féministes, de syndicalistes et de partis politiques progressistes. Alors, pourquoi vouloir le faire entrer dans la Constitution ?

pour exiger de les encadrer, voire de les limiter, surtout lorsqu'il s'agit de la liberté d'avoir ou non un enfant ! Cette situation se retrouve en France, en Europe et dans le monde. En plus de ces blocages idéologiques, j'ai déjà eu l'occasion de décrire, ici même, les embûches matérielles qui entravent le droit à l'avortement dans notre pays

C'est une petite musique que l'on connaît bien et qui présente quelques similitudes avec les années 1970 ! J'espère donc que le Sénat va se saisir, cette fois-ci, de la présente proposition de loi pour consolider ce droit à l'IVG si chèrement acquis. Le constitutionnaliser est une opportunité qu'il faut saisir. En effet, si le Conseil constitutionnel a toujours jugé les lois relatives à l'interruption volontaire de grossesse conformes à la Constitution, il n'a pour autant jamais consacré ce droit sous la forme d'un droit fondamental. Ainsi, l'IVG ne bénéficie que d'une protection législative, et non constitutionnelle. Aujourd'hui, une loi qui porterait atteinte au droit à l'IVG ne serait pas censurée. Mes chers collègues, la volonté de constitutionnaliser le droit à l'avortement n'est pas nouvelle. Elle ne date pas de la décision de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin 2022. Cela fait onze ans, depuis 2012, que le parti communiste porte cette idée le groupe CRCE a déposé une proposition de loi en ce sens dès 2017. Nous le répétons, et comme nous l'avions soutenu récemment lors de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle déposée par notre collègue Mélanie Vogel, dont nous étions cosignataires, il est grand temps de conférer à l'interruption volontaire de grossesse le statut de droit fondamental et de l'inscrire dans la Constitution afin de s'assurer que l'accès à l'IVG ne puisse être affaibli, voire supprimé, par des dispositions législatives.

C'est ainsi que notre collègue Philippe Bas souhaite faire bouger les lignes : il a déposé un amendement qui porte sur l'article 34 de la Constitution, comme le défendait le groupe CRCE.

Mes chers collègues, comme nous y invitent les associations féministes, dont certaines sont ici présentes et que je salue, soyons le premier pays garantissant le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Je fais mien l'appel d'Osez le féminisme ! d'octobre dernier : « Nous appelons la France à être pionnière dans la protection du droit à l'avortement, en devenant le premier pays

sans compter les nombreux textes déposés sur les bureaux respectifs de nos deux assemblées -, une nouvelle proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à

et à l'histoire de chacun et chacune d'entre nous. La genèse de cette multiplication de textes, c'est bien évidemment l'actualité américaine ou plutôt l'actualité d'une juridiction,

du 22 janvier 1973. Ce dernier avait fondé une protection fédérale, sous le contrôle de la Cour suprême, du droit à l'avortement sur le fondement du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis, lequel dispose notamment qu'aucun État « ne privera quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété, sans procédure légale régulière ». Désormais, il appartient à chaque État fédéré américain de légiférer sur l'interdiction ou non du recours à

Comme notre rapporteur nous l'a rappelé en commission des lois, notre arsenal juridique est suffisamment solide concernant l'IVG. En témoigne la loi du 17 janvier 1975 portée par Simone Veil, alors ministre de la santé, relative à Ses dispositions n'ont jamais cessé d'être renforcées par le législateur- allongements successifs des délais, élargissement des praticiens pouvant pratiquer des IVG, etc. -et confortées par le juge constitutionnel. Au-delà de cette intégration pleine et entière dans notre patrimoine juridique, auquel le Sénat est fortement attaché, force est de constater aujourd'hui qu'aucun parti, y compris aux extrêmes de l'échiquier politique, n'a jamais appelé à remettre en cause le principe

dans la Constitution. Avant de constitutionnaliser un tel droit, je pense qu'il est nécessaire de regarder la façon dont il est mis en oeuvre sur le terrain, au quotidien. Malheureusement, à l'heure de la désertification médicale, l'accès à l'IVG est rendu parfois très difficile pour un certain nombre de femmes sur le territoire national.

certains de ses membres soutiendront ce texte, comme ils l'ont fait pour la proposition de loi de Mélanie Vogel, quand d'autres s'abstiendront ou ne prendront pas part au vote, mais la plupart voteront contre l'amendement de Philippe Bas et contre la rédaction issue de l'Assemblée nationale, suivant en cela l'avis de la commission des lois du Sénat.

Lorsque cette thématique est arrivée dans le débat public, j'ai tenté de me poser objectivement les bonnes questions afin d'obtenir des réponses qui dépassent le simple réflexe partisan. Quel est le rôle de la Constitution ? Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est-il en danger dans notre pays ? L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution représente-t-elle une véritable protection supplémentaire dans la défense de ce droit ? Tout d'abord, je pense que le rôle fondamental de la Constitution est de donner la philosophie générale- j'insiste sur ce dernier terme - qui doit présider à la direction de notre pays : forme de l'État, organisation des institutions, règles de production des normes, interactions entre les différents pouvoirs. Je ne crois pas que son rôle soit d'être bavarde, car paradoxalement cela risquerait de l'affaiblir. Si l'on tombe dans un inventaire à la Prévert de l'ensemble des droits auxquels peuvent prétendre nos concitoyens, alors le risque d'insatisfaction permanente nous guette. Nous devons, au contraire, être les garants de la Constitution. Ensuite, je suis toujours étonnée de voir certains débats venus d'outre-Atlantique prendre une place si importante au sein de l'actualité française. Instinctivement, ma philosophie gaulliste m'enjoint de ne point céder aux sirènes de l'actualité court-termiste et je ne peux que regretter ce phénomène de transposition de débats qui n'ont bien souvent pas lieu d'être dans notre pays. Quelqu'un dans cet hémicycle peut-il réellement affirmer que le droit à l'IVG se trouve aujourd'hui menacé dans notre pays ? Peut-on comparer une société où la lutte contre l'IVG est un marqueur politique fort

Enfin, très attachée au droit à l'IVG et à la protection de l'enfant à naître, je me suis imaginé un scénario catastrophe dans lequel une poignée de personnes hostiles à l'interruption volontaire de grossesse prendraient le pouvoir par la force et souhaiteraient abolir ce droit durement acquis. Pensez-vous sérieusement que la Constitution empêcherait quoi que ce soit ? Non, la Constitution ne pourra alors plus rien pour le droit à l'IVG, comme elle ne pourra plus rien pour les libertés publiques, pour la liberté de la presse ou pour la liberté de conscience. Le XX siècle européen est rempli d'exemples de pays qui ont connu un recul des droits fondamentaux à la suite de l'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires. Comment croire que l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution renforcera ce droit ? Je crois que le débat que nous avons aujourd'hui traduit un phénomène bien plus important qui mine le rôle du politique dans notre pays le recul progressif de la capacité à agir sur le réel. Des exemples de combat pour les droits des femmes, il en existe pléthore, et nous savons que, malgré une amélioration considérable de la place des femmes dans notre pays, le chemin est encore long. Nous préférons débattre d'un sujet qui n'en est plus un, certains voient une opportunité de se placer du bon côté du récit, de « faire l'actualité », comme disent les communicants. Mes chers collègues, je pense qu'une partie de la classe politique s'est offert une publicité mépris ! ... mais que cet écran de fumée n'a d'équivalence que l'incapacité à se saisir des thématiques du réel. La posture est facile, faire montre de bons sentiments l'est aussi. Il est bien plus difficile de mener à bien des réformes ambitieuses qui ont un impact sur le quotidien de nos concitoyens. l'éternel débat de la prévalence du fond ou de la forme, mais l'histoire n'est pas dupe. Pour toutes ces raisons et parce que nous croyons à la prévalence du fond sur la forme, le groupe Les Républicains votera dans sa très grande majorité contre cette proposition de loi constitutionnelle. La discussion constitutionnelle. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle

où les femmes sont libres de disposer de leur corps, même si, à cause d'un manque de moyens médicaux, 3 000 à 4 000 Françaises sont forcées de se rendre à l'étranger chaque année, car « hors délais ». Eh oui, l'IVG continue d'être un combat Ce droit concerne également les Françaises vivant à l'étranger. Pour la première fois, le budget 2023 du ministère de l'Europe et des affaires étrangères consacre une ligne budgétaire à nos compatriotes vivant dans des pays où elles n'ont pas accès à l'IVG afin qu'elles puissent la pratiquer en France. Il convient désormais que l'État accélère le déploiement de ce dispositif d'accompagnement, voire de rapatriement, et clarifie les conditions d'accès à ce droit fondamental afin que la protection consulaire inclue l'assistance à l'IVG. Enfin, faut-il rappeler que 81 % des Français sont favorables à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, selon un sondage réalisé en juillet 2022 Alors, mes chers collègues, pour celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus, soyons en phase avec les attentes de nos compatriotes et surtout ne ratons pas l'occasion de confirmer l'exemplarité de la Constitution française en matière de droits fondamentaux et de protection des libertés individuelles.

dont nous débattons ce soir. Ce droit à l'IVG a été inscrit dans la loi grâce à la force de l'engagement d'une femme, Simone Veil, en 1975. Je voterai cette proposition de loi constitutionnelle, comme j'ai voté en faveur du texte de notre collègue Mélanie Vogel à l'automne dernier. J'entends les contestations de mes collègues qui dénoncent l'inscription dans la Constitution d'un droit qui ne serait aujourd'hui pas menacé. Qui peut le certifier ? Pas moi ! J'entends les opposants à l'IVG qui profitent de ce débat pour s'opposer à ce droit, voire qui nous intimident ou nous menacent. Parce que l'IVG doit demeurer un droit fondamental pour les femmes, inscrivons-le dans la Constitution ! Je voterai ce texte, tout en étant consciente qu'il ne constitue pas une fin en soi. Le vote d'aujourd'hui est une étape, un signe envoyé à toutes les femmes et au Gouvernement. N'oublions cependant pas que graver l'IVG dans notre Constitution n'aura de légitimité que si son accès demeure garanti partout sur notre territoire pour toutes les femmes- nous pouvons nous accorder, je le crois, sur cela. Actuellement, il ne l'est toujours pas. Ce vote nous oblige à y remédier au plus vite. C'est un impératif de santé publique face à un délit de non-assistance à femme en danger. Au-delà des rédactions proposées, la question qui nous est posée ce soir, mes chers collègues, est simple : souhaitons-nous

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la question qui nous est posée par ce texte est la suivante : voulons-nous apporter une garantie constitutionnelle au droit à l'interruption volontaire de grossesse ? À titre personnel, je le souhaite et je voterai aujourd'hui, comme en octobre dernier, pour la constitutionnalisation de cette liberté fondamentale pour les femmes. Pourquoi ? Parce que la Constitution est notre texte à valeur suprême ; elle est le socle commun des valeurs et des libertés fondamentales de notre société, celles auxquelles nous ne devons pas déroger. Inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est inscrire ce droit fondamental au sommet de notre hiérarchie des normes, c'est sacraliser un droit qui a fait l'objet de très nombreux combats pour faire partie de notre patrimoine juridique fondamental. À l'heure où les droits des femmes en général et le droit à l'avortement en particulier, peuvent faire l'objet de reculs dans des pays pas si lointains, et même si la situation américaine n'est pas comparable à la nôtre, j'ai la conviction qu'il est pertinent de conférer la plus haute protection à ce droit. Les droits Les droits des femmes nécessitent notre constante vigilance, notre mobilisation et notre action de chaque instant. L'absence actuelle de remise en cause de l'IVG dans notre pays ne saurait nous exonérer de tout faire pour protéger et garantir, dès aujourd'hui, ce droit auquel nous sommes tous attachés.

un événement qui ne nous concerne pas et ne nous regarde pas : une décision de la Cour suprême des États-Unis qui n'a aucun impact sur la France, de la même façon que notre vote n'en aura aucun sur les États-Unis.

Aujourd'hui, j'entends parler de la Constitution comme si c'était un fourre-tout dans lequel nous pourrions inscrire tout ce qui nous tient à coeur, et qui serait alors protégé comme dans un coffre-fort. Là encore, vous savez que c'est faux. La Constitution est l'ensemble des règles qui régissent nos institutions

Or j'entends que certains auraient des positions dignes et d'autres, non. Nous avons toujours des positions dignes dans cet hémicycle ; elles sont diverses, mais elles doivent pouvoir être acceptées. Pour ma part, je ne voterai pas ce texte.

monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne cherche pas à faire durer le débat, mais celui-ci est suffisamment important pour que chacun puisse s'exprimer. Je voudrais faire trois observations rapides.

que ce soit le moment le plus propice pour tenir un débat apaisé sur une question aussi grave que celle-là ? Enfin, troisième observation,

Je voudrais m'adresser à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui pour leur dire que le recours à l'IVG n'est absolument pas remis en cause en France, puisqu'il s'agit de l'un de nos droits fondamentaux. La position constante du Conseil constitutionnel sur ce sujet est extrêmement protectrice. Le recours à l'IVG découle de la liberté de la femme, tirée de l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

à l'IVG. Il n'est pas souhaitable d'attiser des peurs fondées sur la situation d'autres pays. Compte tenu du climat déjà particulièrement anxiogène que connaissent nos concitoyens, il me semble inutile d'en rajouter.

évoquant par une correspondance analogique, formelle, naturelle ou culturelle quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir. Mes chers collègues, en toute honnêteté, que la protection du droit à l'IVG, que je défends de toute mon âme, est absente ou impossible à percevoir ? Le Conseil constitutionnel a, dès 1975, validé la loi sur l'IVG en soulignant que son article 1, qui énonce le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, doit pouvoir connaître des limites- soit, précisément, ce droit à l'IVG que nous revendiquons.

aidera. La parole est à Mme Toine Bourrat, sur l'article. Mes chers collègues, la baisse de confiance accordée par nos concitoyens à la classe politique en général et à l'exécutif en particulier nous oblige. Sans cesse rappelée par les baromètres d'opinion, cette confiance abîmée, qui confine parfois à la défiance, est souvent le fruit des incohérences que nos concitoyens identifient dans les discours tenus par leurs représentants. Elle nous oblige parce que la politique, c'est d'abord des convictions. Nous avons voté contre la constitutionnalisation de l'IVG le 12 octobre 2022 en commission des lois du Sénat. Nous avons voté contre la constitutionnalisation de l'IVG le 19 octobre 2022 en séance publique au Sénat. Nous avons voté contre la constitutionnalisation de l'IVG le 25 janvier 2023 en commission des lois du Sénat. Je ferai donc preuve de cohérence et voterai contre la constitutionnalisation de l'IVG ce soir en séance publique.

chers collègues, je vous le dis comme je le pense : je crois que nous nous fourvoyons. Le mot que nous devrions retenir aujourd'hui et sur lequel nous devons à nos concitoyens de concentrer tous nos efforts est, de mon point de vue, celui d'« effectivité Dire qu'une norme juridique est effective, c'est dire qu'elle existe dans la réalité et qu'elle est appliquée dans les faits. Cette acception classique de l'éminent doyen Carbonnier dans un article précurseur de 1958 renvoie à une application effective effective des normes. Nous sommes favorables à l'effectivité du recours à l'IVG, mais cette effectivité ne se limite pas à l'application d'une règle : elle doit aussi recouvrir une dimension symbolique. Or, comme le doyen Favoreu l'énonçait, si le législateur peut abroger certaines des règles qui protègent ou favorisent l'exercice de droits fondamentaux, il ne pourrait pas le faire au point que ces droits n'aient plus d'effectivité. Dès lors, ne nous trompons pas quant à la question juridique qui nous est posée Faut-il ajouter à notre texte fondamental une disposition déclarative ? Je ne le crois pas, et je n'en ai pas honte, madame Vogel. Ou faut-il agir concrètement en faveur de l'accès effectif de toutes les femmes à l'IVG ?

et une issue hypothétique qui est celle du référendum, les défenseurs de l'IVG imaginent-ils une seconde ce que représenterait un débat sur une question sociétale de cette ampleur dans l'état actuel de la société française ?

je remercie Agnès Canayer, notre rapporteur, de l'avoir bien démontré -n'est menacée en France par aucune formation politique. Le Conseil constitutionnel a, en quelque sorte, constitutionnalisé le droit à l'IVG,

Enfin, est-il raisonnable de vouloir constitutionnaliser à tout va ? Dominique de Legge l'a très bien dit, ce pourrait être demain, par exemple, le droit au suicide assisté ou la PMA pour toutes. Pourquoi ces droits

la constitutionnalisation du droit à l'IVG est inutile et dangereuse. Elle est inutile, car il n'y a pas de sujet chez nous en France : le droit à l'IVG n'est pas menacé. Alors pourquoi cette proposition ? Pourquoi cette obsession de la gauche ? La principale raison en est la frustration,

Merci,

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.